La séance est reprise nous reprenons la discussion de la proposition de loi visant à protéger les logements contre l'occupation illicite, nous poursuivons la discussion générale. Et nous sommes parvenus à l'intervention de Monsieur Dominique Théophile qui a la parole pour ces 4 minutes.

Monsieur le président. Monsieur le Ministre, chers collègues. Nous sommes aujourd'hui réunis pour examiner une proposition de loi très attendu. Comme vous monsieur le rapporteur. Nous considérons que le texte adopté par l'Assemblée nationale en 2ème lecture constitue un bon compromis. Il permet en effet de lutter plus efficacement contre le squat tout en améliorant l'accompagnement des locataires en difficulté. Il permet également d'assurer un équilibre entre la défense du droit de propriété et la protection du doigt au logement. Le durcissement des peines encourues en cas de violation de domicile. La création de délit d'occupation frauduleuse. D'un local ne constituant pas un tout. Un domicile. La répression de la propagande et de la publicité en faveur. Du squat et l'alourdissement des peines applicables aux marchands de sommeil sont autant de réponses concrètes aux situations dramatiques et traumatisante auquel sont aujourd'hui confrontés, nombre de nos concitoyens. Plus largement. C'est la santé économique du secteur du logement, qu'il s'en trouvera améliorée. Les mesures prévues par la proposition de loi sont en effet de nature à rassurer le bailleur des bailleurs quant à la sécurité de leur investissement. Nous constatons avec satisfaction que le texte soumis à notre examen comprend de nombreuses dispositions issues d'amendements sénatoriaux. Mes collègues du groupe RDPI et moi-même sommes heureux d'avoir pu contribuer à l'amélioration du dispositif proposé par l'Assemblée nationale. À cet égard nous nous réjouissons que nos collègues députés est maintenu à l'article 1er à. La disposition issue d'un amendement du président Patriat qui prévoit une gradation entre la peine prévue pour le squat de domicile et celles applicables aux squat de locaux ne constituant pas un en ce qui concerne l'article 1er s'est je salue la sagesse de nos collègues députés qui ont supprimé la disposition qui tendait à obliger le préfet de département à appliquer une décision d'expulsion rendue par le juge dans un délai de 7 jours. Cette disposition risquait de porter atteinte au droit au recours aussi. Elle aurait sans nul doute été censuré par le Conseil constitutionnel. Vous l'avez dit monsieur le rapporteur. Depuis l'adoption du texte en première lecture par le Sénat. Le Conseil constitutionnel a jugé conforme à la Constitution la procédure accélérée d'expulsion que l'article 2 de la proposition de loi prévoit d'étendre aux locaux à usage d'habitation. Tirant les conséquences de la réserve d'interprétation formulées par les sages de la rue Montpensier. L'Assemblée nationale a opportunément introduit une disposition prévoyant l'obligation par le préfet de prendre en considération la situation personnelle et familiale du squatteur. Préalablement à la mise en demeure de quitter le logement. Nous saluons cette excellente initiative qui permet de sécuriser juridiquement le dispositif s'agissant de l'article de terre. Nous nous félicitons du renforcement du contrôle de la mise en oeuvre du dispositif de mise à disposition temporaire de locaux vacants à des fins sociales l'État aura ainsi la possibilité de prévenir tout risque de voir des entreprises se saisir du dispositif à des fins contraires à son objet social. Mes chers collègues comme moi vous avez peut-être entendu parler de ce terrible drame. grande colombe ah Garenne-Colombes le 3 juin dernier. Une sexagénaire ayant accumulé d'importantes dettes de loyers auprès d'un bailleur social cette S'immoler devant la mairie. Cette personne a malheureusement succombé à ses blessures. Cette situation tragique montre combien il est urgent de renforcer l'accompagnement des locataires en difficulté. Telle est l'objet des articles 5. 7 et 8 que l'Assemblée nationale a adopté conforme lors de la deuxième lecture je conclurai mon propos en remerciant au nom du groupe RDPI le président Kasbarian au groupe Renaissance et Horizons de l'Assemblée nationale qui nous ont permis de prendre à bras le corps la problématique du squat et du contentieux locatifs bien évidemment le groupe RDPI votera le texte. Merci cher collègue. Et la paix. À présent, la parole est à monsieur Denis Bois-d'de pour le groupe socialiste, écologiste et républicain, et il a six minutes. Merci monsieur le président. Messieurs les ministres. Monsieur le rapporteur, chers collègues. On dénombre en France 4,15 millions de personnes mal le vote la loger. Ce sont là les chiffres du dernier rapport annuel de la Fondation Abbé Pierre publié le lendemain de l'examen de ce texte en première lecture par notre assemblée. dit qu'on utilise cette proposition de loi dite anti-squats. On pourrait être tenté de mettre ce chiffre en comparaison avec les 5, 42. Situation de squats recensés chaque année dans le pays. Mais cela me semble pas pertinent. Ce ne serait pas pertinent, car ce texte mal de renommé de se concentre pas uniquement sur les questions de quoi le squat mais il vise également les locataires en difficulté qui se trouve en situation d'impayés. Dans le contexte actuel légiférer sur l'enjeu central de l'autre à travers une très la proposition de loi nous semble symbolique d'une certaine forme d'aveuglement vis-à-vis de l'actuelle crise de logement et ses conséquences dans le pays. La construction de logements sociaux. La lutte contre la vacance. La revalorisation des aides au logement, la rénovation de technique thermiques massives. Aux yeux de Sonia sur sénateur socialiste. Il existe tellement de. Qui semblaient prioritaires et pour l'écrire des réponses gouvernementales ne sont pas à la hauteur. C'est pour porter ses ambitions. Monsieur le Ministre que dès septembre 2002. Nous avions appelé à faire appeler à faire du logement. La grande cause nationale de ce quinquennat. Malheureusement ce texte qui nous vient de l'Assemblée nationale porte une ambition. Ne différentes. Si nous sommes convaincus de la nécessité de protéger les propriétaires contre des situations abusives. Il nous semble essentiel de préserver l'équilibre comme vous l'avez dit, monsieur le ministre, entre le droit à la propriété et le droit au logement. Or cette proposition de loi vient rompre cet équilibre qui compte. Il a été construit au travers des différentes décennies sans pour autant apporter de nouvelles garanties concrètes aux propriétaires. En tant que législateurs, nous devons être attentifs à l'efficacité des dispositifs que l'on propose. À ce titre, on peut s'interroger sur l'intérêt de la création d'un délit sanctionnable amende à 7500 euros pour le locataire. Un défaut de paiement qui se maintiendrait dans le logement. cette mesure n'apporte strictement rien aucune plus Value au propriétaire. Ce ne sont pas eux les bénéficiaires de 7500 euros et nous savons d'ailleurs que dans la plus grande majorité des cas les dettes locatives ne sont pas récupéré par les propriétaires. Il en sera de même évidemment pour le recouvrement de cette amende. En effet, rares sont les locataires qui choisissent de ne pas payer leur loyer, de se retrouver en situation d'expulsion. Au final, cet article aura pour seule conséquence l'engorgement notre appareil judiciaire. En première lecture nous avions également dénoncé la réduction des délais entre le commandement à payer et l'assignation à la justice. De l'avis de la vie des professionnels comme des associatifs, cette période est essentielle. Pour mener tout le travail d'accompagnement social nécessaire dans le cadre, une procédure d'expulsion. C'est d'ailleurs ce travail qui dans certains cas permettra de trouver des solutions de paiement qui serait profitable aux 2 parties. Alors oui, on peut avoir une discussion sur la durée des procédures de la solution. Allô dure en moyenne entre 18 et 24 mois du lancement de la procédure à l'expulsion définitive en comprendre. Disons que l'enjeu n'est pas de réduire de 15 jours entre le délai de commandement demain et l'assignation. Non, dans un grand nombre de cas, la presse IKEA le code de l'allongement de la procédure réside dans l'absence de solution de relogement. cette absence de solution de relogement qui empêche. Le concours de la force publique. Le difficile au relogement des locataires menacés d'institutions est aujourd'hui renforcée par la pénurie de logements sociaux.

En contribuera moment fragilisé le secteur de logements sociaux. Les bailleurs sociaux n'plus aujourd'hui la capacité de produire dedans pour de logement suffisant. La construction de logements sociaux a chuté de 40%. Entre 2017 2022 ce 115 milliards d'euros d'économies qui ont été réalisées sur le logement des Français les plus modestes. Malgré de nombreux signaux d'alerte. Le mois dernier le Ministre des comptes, des comptes publics, annoncé que le ministère du Logement seraient particulièrement concernés par la baisse des dépenses publiques envisagées sur le budget 2024 alors. Alors après la baisse des APL. Après les milliards d'euros d'économies sur la RLS. Que sera la nouvelle baisse de crédits des politiques du logement. Et surtout, quelles seront les conséquences pour les Français qui ont dans de plus en plus de mal à se loger. Cette proposition de loi ne résout pas le problème des propriétaires. Mais elle pourrait accélérer la après que Brigitte a après que précarisation extrême de certains locataires. Les acteurs associatifs mais aussi le défenseur des droits, et même le rapporteur spécial de l'ONU en charge du logement et de l'extrême propreté ce sont côté des des conséquences de cette proposition de loi. Ce dernier dans un courrier adressé au gouvernement en alerte et l'absence d'étude d'impact sur les conséquences qui pourraient résulter des changements introduits dans ce texte. Messieurs les ministres. Nous pensons que ces questions devrait vous interpeller. C'est pourquoi une nouvelle fois les sénateur socialiste, écologiste et républicain s'opposeront à cette proposition de loi. Merci. Très bien, chers collègues. À présent, la parole est à madame Marie-Noëlle Lienemann pour 4 minutes. Et pour le groupe CRCE. Messieurs les Ministres, Monsieur le Président, messieurs les rapporteurs, chers collègues. En première lecture, nous avons déjà dit tout le mal qu'on pensait de cette loi. Et nous avons voté contre. nos arguments pouvait se résumer en quelques phrases. Cette loi déséquilibre des rapports entre propriétaires et locataires au détriment des locataires et plus généralement fragilise davantage. Les familles les plus démunies et les mal logés. Au motif de traiter un nombre infime. De situations où des petits propriétaires leur domicile squatter chez eux là où ils vivent. Et qui effectivement déjà dans la loi il y a des outils, mais mérite peut être encore un durcissement. Mais c'est une part infime. Vous avez utilisé ces faits divers et ces drames pour justifier une loi qui est en fait. Une une offensive contre les les locataires et une offensive contre les plus démunis. Les arguments que nous avions donné alors sont encore plus fort aujourd'hui hélas parce que la situation s'est détériorée. En première lecture, nous disions déjà que il devrait pas y avoir d'expulsion sans relogement. c'est parce que le logement n'est pas un bien comme les autres, c'est un élément essentiel de la dignité humaine et que quand on expulse quelqu'un, quel que soit le statut dans lequel il était auparavant le mettre à la rue n'est pas une solution, d'autant que je rappelle que le président de la République avait dit en 2017 qu'une de ses priorités, c'est qu'il y ait plus personne à la rue, aujourd'hui. Rod politique en mai davantage. Deuxièmement, nous disions que la meilleure solution c'est d'en, d'avoir une politique. Plus favorable à la mise en oeuvre du Dalo du logement d'abord du droit au logement pour tous des cons des des outils pour mieux combattre les impayés. Je vous rappelle que nous avons toujours défendu la garantie universelle des loyers qui avait été voté lors de la loi allure au Sénat et qui garantirait de manière équilibrée, les propriétaires elle les locataires et de l'autre côté, nos institutions sur la revalorisation des APL pour limiter les impayés. Que voyons-nous depuis. Le nombre d'impayés. Monde de manière extrêmement préoccupante. C'est récent. C'est vrai qu'après le Covid, on n'avait pas eu ce mouvement on là maintenant de manière très importante, sans doute la conséquence de l'inflation. Le deuxièmement le nombre de demandeurs de logements HLM a connu un bond considérable. Troisièmement. Nous voyons aussi que. Les les APL ne couvre pas l'essentiel des dépenses de logement des familles modestes, notamment au regard de l'augmentation de la quittance et des charges. Alors là vous êtes en train de nous faire le en même temps. Le en même temps, c'est en même temps que durcit les lois en direction des locataires et des plus démunis et en même temps on prend pas les décisions qu'il faut pour contrecarrer la crise du logement, puisque les conclusions du CNR logement ne peuvent que nous inquiéter quand tu as ça dit aux décisions prises. Je prends plusieurs exemples. Padraig pas de de régulation des loyers. assez à 3,5 mais la fonction publique de 1 5, c'est-à-dire ça ne suit pas l'évolution de l'inflation. Pas d'augmentation des aides à la Pierre, pas de baisse de la TVA. Pas de remise en cause de la ARS et même pour le logement d'abord qui devrait être une des cibles par rapport au sujet que nous traitons vous proposer simplement 160 millions d'euros supplémentaires alors que les associations mettaient leur seuil minimal c'était les conclusions du CNR à 400 millions d'euros. Bref, la politique que vous menez ne va faire qu'accroître les problèmes menace dans certains cas la dignité d'un certain nombre de nos concitoyens ne résoudra en réalité aucun des gros problèmes. Et notamment des cas marginaux qui pouvaient être traités nous êtes nous maintient notre vote contre cette loi et je voudrais vous dire Monsieur le Ministre. Je, j'ai été meurtri

que dans les impayés de loyers. Dans les dans les champs qui squattent, vous l'avez dit, monsieur le Ministre, vous avez parlé de je défends les honnêtes gens, il y a des gens qui sont tout à fait honnête mais en détresse sociale de la même manière. Oui, nous ne sommes pas pour la politique des squats. Nous sommes pour la politique qui garantit le droit au logement plus démunis contre les squats. La parole est à présent Madame Goulet. Pour le groupe de l'Union centriste et la six minutes.

Je ne comprends pas qu'il reste encore autant de manichéisme dans ce texte avec d'un côté les gentils. Protecteur des mal logés et de l'autre côté les méchants défenseur des propriétaires, ce texte ne mérite pas tant d'indignité. Il n'est pas destiné à régler l'ensemble des problèmes du logement. Il est destiné à régler le problème du squat, je pense qu'il y a un objet très déterminé et je crois que ce texte fait bien de le régler. Le fait d'être mal logés ne justifie pas évidemment le squat. Le fait d'être propriétaire ne protège pas difficultés financières et il serait temps donc de sortir de ce manichéisme. Le présent texte port sur l'occupation illicite des logements qui recouvre à la fois le phénomène du squat et celui des locataires défaillants. On distingue évidemment bien les deux et il faut rendre hommage au rapporteur André Reichardt a Dominique Estrosi Sassone à Madame, Létard et aussi à Noëlle Lienemann qui sont dans cette maison. Les bonnes fées du droit au logement et de l'urbanisme. Leur travail, celui de la commission des lois et des affaires économiques a permis de rééquilibrer un texte qui n'était pas aussi équilibré après sa première lecture au Sénat. Je voudrais faire quand même une petite parenthèse. Monsieur le Ministre de lecture sur un texte, un texte non en urgence a quand même beaucoup d'avantages. Ça évite, probablement des malfaçons et ça permet quand même dans un délai raisonnable de voter des textes qui sont d'un peu de meilleure facture que des textes qui sont votés. Au lance-pierres. Nous avons des squatters sans droit ni titre qui élève par moment la violence de domicile au rang de combat idéologique utilisant notamment le guide du squat pour lequel évidemment, nous avons pris des dispositions concernant sa publication les propriétaires comme les locataires peuvent être victimes de squat, on a des chiffres. Nous avons aussi souhaité renforcer la lutte contre ce phénomène en supprimant la possibilité pour le juge d'accorder des délais un squatteur faisant l'objet d'une décision d'expulsion. En cela, nous envoyons un signal clair à ceux et celles qui pensent pouvoir ignorer le droit de propriété consacrés par la déclaration des droits de l'homme et du citoyen d'un autre côté nous avons des locataires qui ne payent pas, ou plus leur loyer le texte dans ce cas fait bien la différence entre les accidents de vie et les locataires de mauvaise foi. C'est là que la présence du garde des Sceaux a toute sa. Son intérêt parce que les commandements de payer qui sont adressées et qui sont éventuellement défaillant. Vous avez ici un binôme avec le ministre en charge du logement. Tout à fait efficace et comme on vient de voter un texte sur la justice. En même temps. Ça me semble une bonne idée, que vous soyez tous les deux au banc aujourd'hui pour pouvoir régler les problèmes qui, d'une façon ou d'une autre se régleront aussi au moment du projet de loi de finances. Parce que là aussi il va falloir assurer les moyens d'exécuter ces décisions. Donc les locataires défaillants ne doivent pas être mis sur le même plan que les locataires défaillants de mauvaise foi et encore moins que les squatteurs. C'est pourquoi nous avons tenu au Sénat à maintenir les pouvoirs d'office du juge pour l'octroi de délais de paiement aux locataires de bonne foi, donc ce n'est pas non plus un texte. d'autres locataires de mauvaise foi qui refuse de régulariser leur situation, de quitter leur logement. De manière illicite son eux pénaliser c'est l'équilibre que le Sénat et l'Assemblée nationale ont trouvé. Le texte tel qu'il ressort de l'Assemblée nationale et du travail au Sénat. Rempli sa fonction, c'est-à-dire la lutte contre les squats en alliant ses considérations d'efficacité et de justice, nous semble-t-il. Nous parviendront ainsi à rétablir la confiance des Français dans la propriété. Il est vrai que ces squats sont des mesures et des opérations extrêmement irritante qui font certes la première page des journaux qui sont peut être des opérations marginal mais qu'il convient de régler. C'est l'objectif de cette loi, elle est atteinte et nous voterons ce texte je vous remercie de votre attention. Monsieur le président. Monsieur le Ministre. Sur le rapporteur, chers collègues. La conception qu'ont nos sociétés de leur propriété le régime juridique qui lui est associé sont parmi les éléments fondamentaux de notre droit de Luca Russo. L'idée de propriété a su mobiliser de nombreux auteurs tout au long du. Chez Hackl. Et dans les traces des débats se retrouvent dans nos textes fondateurs tels que la déclaration des droits de l'homme, qui souligne. Je me permets de le rappeler que le but de toute façon je suis un homme politique. Est la conservation des droits naturels imprescriptibles de l'homme, parmi lesquelles la liberté la propriété. Aux législateurs d'agir pour éviter que des propriétaires se retrouvent désemparés. Face à l'occupation de bien qui a nécessité parfois des années de travail de sacrifice. Chacun a en tête les affaires médiatisées de personnes retraités à faibles revenus. Dans les résidences se retrouve squatter et pour les cas le l'administration ne semble impuissante à réagir. Bien sûr. Dire qu'il faut défendre les propriétaires ne signifie pas que nous ayons pas conscients et c'était réalité sociale qui conduisent à ces situations dramatiques. La précarité la paupérisation dans notre société doivent être combattus en même temps qu'il faut garantir le respect de la propriété. C'est être naïf de le rappeler. Mais l'État français devrait être en mesure d'un côté, de protéger les occupations, ville du site. Et de notre de veiller à la prise en charge des personnes démunies. Nous constatons hélas. Qu'il y a des de faïence. Sur ces 2 sujets. Quoi qu'il arrive le soir sur cette question de la répression du squat. Cette proposition de loi est donc la bienvenue. Je pense en particulier aux dispositions pénales. Introduite par ce texte et qui combler une lacune de notre droit. Car comment imaginer. Il n'existe à ce jour ni délit ni peine pesant sur l'occupation d'un immeuble au Sun titre sur le fond seul de la tête trop droit de propriété, indépendamment de la notion de domicile. Et ce. Ironie du calendrier de l'agenda du Sénat. Quelques jours après avoir examiné le projet de loi sur la douane qui mettait en avant cette notion de domicile. Il faut que la loi incrimine ces ajustements largement et les cantons de peine me semble juste. Toutefois, nous saluons les apports du Sénat sur cette nouveauté. Qui permettront de parfaitement distinguer le squatteur du locataire pour ne sanctionner que le 1er des 2. Nous sommes également favorables à à la nouvelle prorogation par l'article de but du dispositif. Qui avait déjà introduit la loi du 20 seule, De mobilisation pour le logement et la lutte contre l'âge. Locale, ouvrait la possibilité de confier à des organismes agréés. L'occupation temporaire de locaux vacants afin d'assurer leur protection alors près la Car naturellement abordé le problème des occupations ville du shit c'est aborder aussi celui des locaux vacants, notamment dans les zones hyper urbanisée au regard des problèmes de logement social. Concernant le second volet de ce texte, nous avons été partie que vigilant. Chorus Fernand les dispositions portant sur les locataires en difficulté. Nous ne souhaitons pas qu'on a le me soit fait entre 2 situations fondamentale différente. Celle des squatters et celle des locataires en difficulté. Dès la première lecture notre groupe s'était inquiété d'un possible le déséquilibre. Entre les droits des propriétaires et la protection des locataires. Toutefois le texte. Tel qu'il vous est présenté à l'issue de la navette semble. Satisfaisant et non c'est sûr Constance. Comme lors de leur première lecture nous voterons en majorité au sein du groupe RDSE en faveur de cette proposition de loi. Je vous remercie. Monsieur le président, monsieur le garde des Sceaux, Monsieur le Ministre du Logement. Monsieur le président de la commission de lois. Monsieur le rapporteur. Mes chers collègues. Avec cette seconde lecture. Nous arrivons au terme de l'examen de cette proposition de loi qui ne contient que quatre article en débat la plupart ayant d'ores et déjà été votée par l'Assemblée nationale dans leur rédaction établi par le Sénat. Je tiens tout particulièrement à remercier le rapporteur André Reichardt avec qui nous avons pu travailler de façon très constructive, tant lors de la première lecture que tout au long de la navette. Je voudrais rappeler ce soir l'apport important du sénat dans ce texte et faire deux observations sur les dispositions restant en discussion d'abord rappelé les apports majeurs du Sénat concernant la répression du squat et la gestion des impayés de loyer le squat est un viol de l'intimité et nous souhaitons qu'il soient réprimer sans faiblesse, je me réjouis donc que ce texte est permis d'y intégrer l'essentiel des dispositions de la proposition de loi que j'avais déposée et qui avait été votée en janvier 2020 par le Sénat. Il sera désormais possible de s'attaquer aux réseaux qui organisent et favorise le squat la protection du domicile était tendue en outre en pérennisant le logement intérimaire sous contrôle strict de l'État on promeut une alternative légale à l'occupation de sites inoccupés au bénéfice de personnes fragiles ou en mobilité. Concernant les impayés de loyers. La porte du Sénat a également été déterminant dans l'intérêt des propriétaires, comme des locataires. Nous avons préservé les possibilités d'un accord amiable et d'un règlement de la dette locative sous l'égide du juge qui doit pouvoir vérifier le montant de la dette et la décence du logement mais également établir un échéancier et des délais de paiement sur la base d'un diagnostic social et financier renouvelé sur ma proposition. Le Sénat à renforcer l'accompagnement des locataires en difficulté et la prévention précoce des impayés et des expulsions dans un nouveau chapitre de la proposition de loi qui a été et je m'en réjouis, définitivement adoptée par l'Assemblée nationale. Dans chacun de nos départements. La saisine des commissions de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, les fameuses CAPEX se fera donc beaucoup plus tôt et elles auront des pouvoirs renforcés en outre le temps disponible pour la réalisation du diagnostic social et financier sera doublé, il en résultera ainsi une dette, amélioration de l'action des travailleurs sociaux dans les dispositions qui sont encore en discussion. Je voudrais relever 2 points le 1er et que le texte a pu être adapté et sécurisé pour tenir compte de la récente décision du Conseil constitutionnel validant la procédure d'évacuation forcée prévue par l'article 38 de la loi Dalo, notamment lorsque le logement squatté et le futur domicile de la victime notamment lorsqu'elle vient de l'acheter ou de conclure un bail. Le second point concerne la procédure d'impayés. Il conviendra que le préfet informe des locataires de l'ensemble de leurs droits en matière de délais de paiement, mais aussi de maintien dans les lieux cet élément sera également essentiel dans la réforme du diagnostic social et financier qui résultera de ce texte, il est en effet de l'intérêt des deux parties que ces 2 éléments aillent de Pair, afin que le locataire conserve son logement et que le propriétaire récupère son dû. Il n'y aurait pas de sens à ce que le juge met en place un échéancier sans le corollaire du maintien dans les lieux ainsi. Je pense que nous avons pu trouver un équilibre en étant plus ferme contre les squatteurs et les locataires de mauvaise foi, tout en assurant une meilleure prévention des expulsions, sans en faire porter le poids sur les propriétaires. C'est la raison pour laquelle le groupe Les Républicains votera cette proposition de loi. Merci cher collègue. La parole est à présent à monsieur Pierre mais de vielles pour les indépendants.

Monsieur le président. Monsieur le garde des Sceaux, Monsieur le Ministre, monsieur le président de la commission des lois. Monsieur le rapporteur. Mes chers collègues. En France, défendre au Louvre droits de propriété. N'est pas toujours chose aisée. C'est un comble au pays des droits de l'homme. Car ce droit rappelons-le y occupe une place centrale dans la déclaration de 1789. Il est figure en 2ème position de la liste établie par l'article de. Juste après la liberté. Et excusez du peu. La sûreté et la résistance à l'oppression. Défendant le droit de propriété. Ce n'est pas prendre parti pour les propriétaires. Ce n'est pas ignorer les difficultés sociales. Ce n'est pas non plus milité contre le droit au logement. C'est simplement des formes de la démocratie et ses valeurs. Il me paraît important de rappeler ces évidences. Car le droit de propriété et de plus en plus malmenés en France de facto et de jurer. De facto, parce que les intrusions et occupations illicites sont devenus chose commune. Et ce, dans l'ensemble du territoire national. Nous avons tous en tête des affaires de familles de couples de personnes âgées soudain privés de leur logement par des squatters. Il se retrouvent du jour au lendemain dans une situation extrêmement difficile. À la fois obligé d'assumer les charges induites par le logement dont ils ne jouissent plus. Et privé d'ambiance qui leur est cher. Surtout face à la complexité juridique et administrative. Ces personnes qui voient leurs droits bafoués. Pensent que la situation profite à ceux qui ont enfreint la loi. Et qui ne sont pas tenus de rendre des comptes. Cette situation donne à penser qu'il existe une impunité pour ceux qui ne respectent respectent Il y a là un terreau fertile de réaction très virulente chez ne s'exprime pas dans les faits. Ces réactions ne s'exprimeront dans les urnes. Car et c'est mon second point. Le droit de propriété est aussi malmenée de jurés. Nos propres textes de loi ont tendance à protéger les locataires contre les propriétaires. La tendance n'est pas nouvelle. Arthur Levasseur Premier Ministre du logement de France en responsabilité lors du Cartel des gauches déclaré devant la Chambre des députés. Je serai le ministre des locataires. Depuis lors. Notre droit n'a cessé de mieux protéger les locataires. Pour contrebalancer le pouvoir dans les propriétaires disposent de fait. Ce rééquilibrage. Dans la mesure où il permet d'éviter que des foyers précaires ne se retrouvent à la rue. Mais les abus sont désormais légion. Et relève le plus souvent de la mauvaise foi ou de la malhonnêteté que de la précarité. C'est pourquoi il était nécessaire de redonner force à la justice pour lutter contre l'occupation illicite des logements. Cette proposition de loi est la bienvenue. Je me réjouis que le Sénat puisse l'adopter aujourd'hui sans modification afin de faciliter sa mise en oeuvre rapide. L'Assemblée nationale en 2ème. Lecture à conserver la plupart des améliorations que le Sénat avait apporté en première lecture. La réduction des délais, la simplification des procédures et l'aggravation des sanctions contre les squatteurs sont autant de réponses que nos compatriotes attendent depuis longtemps. Enfin. Le chapitre 3 de la proposition de loi qui vise à mieux accompagner le locataire en difficulté permet d'équilibrer le dispositif est d'apporter une réponse certes incomplète. Mais effective face à la crise du logement qui s'annonce. Comme lors de la première lecture notre groupe votera à l'unanimité ce texte. Merci, cher collègue, la parole est à présent à Guy Bénard Roche pour le groupe écologiste solidarité et territoires et également pour 4 minutes. Bon voilà. Monsieur le président. Monsieur le Ministre. Sur le rapporteur, chers collègues. Deuxième lecture d'une PPL discutable. Qui est censé porter sur le sujet sensible est primordial du logement. Discutable car le titre est trompeur puisque le logement n'est pas le sujet central de textes qui se focalise en fait sur un amalgame entre le logement le domicile et la propriété. Au delà. De dérive certaines qui qui était due à la précipitation dans l'écriture lors de la première lecture que le Sénat avait atténué d'ailleurs. Dans sa grande sagesse cette PPL est basée sur une prémisse très simple le squat seraient la conséquence de la carence du droit actuel insuffisant à dissuader les squatteurs et leurs complices entre guillemets et à garantir le droit des propriétaires il présuppose d'une manière que je trouve caricatural. Une absence d'équilibre qui prétend corriger entre le droit au logement et le droit à la propriété. Dans la réalité, la résolution de ces cas certains très médiatique a permis de démontrer que le droit des aujourd'hui permet déjà ces résolutions sans besoin de modifications législatives. Bien sûr qu'il faut permettre aux coureurs rapide à l'autorité publique pour expulser des occupants des occupants illégaux de domicile principal ou secondaire et la loi ASAP adopté ici aussi en octobre 2020 le permet et a même considérablement durci déjà la répression à l'écart des occupants. Pourtant les auteurs de cette PPL propose d'aller plus loin. Moi je dirais beaucoup trop loin. L'émotion, l'emballement médiatique sur des opportunités pour permettre à certains de prôner une répression sévère sans différencier par exemple les locaux occupés ou pas ou l'état de ces locaux. Je rappelle que la notion de domicile et sa protection relève principalement du droit à la vie privée. Le texte à l'étude souhaiterait étendre et infliger de nouvelles sanctions à toutes les personnes qui se battent dans un bien immobilier, quel que soit son d'usage et quelle que soit sa vacances. Appliquer ce texte à la lettre pourrait doubler le nombre de personnes sur domicile c'est ce qu'a dit le Secours catholique, le texte représente une régression rare du droit au logement, d'après cette même association et d'inquiétantes criminalisation. La défenseure des droits, d'où la rappeler en audition aujourd'hui de la pauvreté. Ce qu'il dit, si cette loi, ce sont bien des délits d'introduction et d'occupation de biens immobiliers basée non plus sur le domicile mais sur le fait que ce bien serve de logement. À l'heure où tous, constate l'échec du CNR, monsieur le ministre du Logement sur une simple vision de la problématique du mal-logement reste un sujet majeur. 3,9 millions de mal logés dans notre pays 300.000 SDF qui est pourtant pas abordé ni même pris en Côte dans ce texte pourtant 2000 va de avant le passage de cette loi, 17.500 ménages ont été contraintes quitter leur logement, avec le concours de la force publique. Il s'agit déjà du plus haut niveau d'expulsions locatives jamais enregistré. Le droit au logement est reconnu comme objectif de valeur constitutionnelle. Les politiques du logement en France dans pas réussi à prendre en compte ce principe. Alors renforcer l'arsenal pénal en étendant en quelque sorte le chant des squatters et le périmètre des condamnés possible dans ce contexte d'expansion du mal logement nous paraît au mieux inappropriée. Enfin ce texte, je le souligne a pas bénéficié du d'étude d'Pâques la majorité présidentielle ayant préféré la proposition de loi au projet de loi ce qui est regrettable. Les carences de l'État, couplée aux dispositions de ce texte ou de trop grande possibilité de sanctions non pas lié à une situation de squat à tolérable mais à des occupations en lien avec des actions revendicatives militante voire des réquisitions légitime. L'occupation illicite par des associations ou des collectifs de bureaux vides depuis des années. Pourra-t-elle être sanctionnés. Oui. Qu'en sera-t-il des pénalités encourues pour l'occupation du de réception d'une entreprise lors d'une action associative ou militante. La loi pourrait-elle s'appliquer à l'occupation de terrain sans destination de local agricole non explicitée sans meubles. Oui, les propriétaires de peuvent plus subir les défaillances de l'État est capable parfois lorsqu'ils sont dans leur droit de leur permettent de reprendre possession de leur logement. Je conclus Monsieur le Président. Nos préoccupations sur les conséquences de ce texte à un moment où l'accès au logement devient un problème majeur dans d'autres pays amène le groupe écologiste solidarité et territoires à s'opposer à cette à ce Le dernier orateur et notre collègue Jean-Claude. Pour le groupe des Républicains. Et il dispose de cinq minutes. Monsieur le président, monsieur le garde des Sceaux, Monsieur le Ministre. Monsieur le président de la commission des lois. Monsieur le rapporteur. Mes chers collègues. Après une première lecture au Sénat en décembre 2022, la navette parlementaire permet aujourd'hui la poursuite de l'examen de cette proposition de loi. Cette proposition de loi visant à protéger le logement contre l'occupation illicite et la démonstration que l'examen parlementaire. Est un facteur d'amélioration des textes, des textes à condition de laisser au Parlement le temps de travailler lors de la navette parlementaire chaque chambre a pu enrichir le texte, jusqu'à arriver un texte permettant un vote conforme. L'atteinte à la propriété privée est un problème public d'ampleur et ça a été rappelé toute la soirée 500.000 commandement de payer et 150.000 assignation en justice pour 70.000 décisions d'expulsions ferme dont 16.000 nécessitant le concours de la force publique. Ce texte dispose d'une forte dimension symbolique. En ne laissant plus organiser un état de fait d'occupation illégale de propriété privée ou de loyers impayés ce texte permettra de renforcer la confiance dans l'État et les pouvoirs publics. Dans un souci de justice ce texte défend avec équité que la loi soit appliquée, et qu'une personne ne puisse se retrouver abusé impudent impunément de c'est bien. Cette proposition de loi là donc pas. N'a dit donc pas une réponse de plus à un fait divers. Il s'agit d'un texte avec une portée certaines sur un enjeu majeur dont on ne peut dont on peut regretter que la politisation et empêcher d'avancer précédemment sur le sujet. Cette proposition s'inscrit en effet à la suite de plusieurs travaux sénatoriaux en particulier avec la proposition de loi déposée par notre collègue Dominique Estrosi Sassone et adopté par le Sénat en janvier 2020 et dont je salue ici le travail conséquent engagé sur le sujet. Le texte vise à mieux protéger la propriété privée quand tous les squatters, ce qui est un droit inviolable et sacrée, selon l'article 17 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Le texte vise également à rééquilibrer les rapports locatifs, à la lumière de nombreuses difficultés rencontrées par les propriétaires confrontés aux impayés de loyers. Il s'agit d'un texte qui va permettre de rassurer les propriétaires et de favoriser on peut l'espérer le maintien et la mise en location de biens dans un contexte de très forte tension dans le secteur immobilier. À la suite de récentes contrainte subie par les propriétaires avec notamment la rénovation énergétique et la fixation des loyers. En première lecture, la commission des lois et la commission des affaires économiques du Sénat ont réalisé. Cela a été rappelé un travail conséquent avec l'adoption de 28 amendement permettant notamment de distinguer la situation du squatteur de celle du locataire défaillant et de prévenir est-ce expulsions locatives dans l'intérêt commun des propriétaires et les locataires. Le texte permet également d'une part d'améliorer l'application de la loi particulièrement difficile en matière d'occupation illicite, logement et, d'autre part d'accélérer la procédure contentieuse. Je terminerai mon intervention avec une pensée particulière pour les maires confrontés à ce type de problème de logement, il recueille les doléances de leurs administrés et en tant qu'élu de proximité, ils sont les premiers confrontés aux tensions. Résultat de ces situations. Il faut espérer que les, les élus locaux constateront que la situation s'améliore. Après ce texte. Enfin je mentionnerai les préfets qui sont les acteurs, des acteurs essentiels du sujet par chargé d'exécuter les décisions de justice avec le recours à la force publique. Il s'agit de décisions forcément difficile mais aussi nécessaires à l'application de la loi dont nous souhaitons tous qu'elle soit plus efficace. Je vous remercie. Merci, chers collègues, la discussion générale est Close. Nous devons passer à la discussion de la motion tendant à opposer luxe exclure du. De d'irrecevabilité. En effet, Monsieur Pascal Savoldelli et les collègues de son groupe ont déposer une telle motion distribuée sous le numéro 5 et à opposer l'exception d'irrecevabilité au texte, en discussion. Pour la soutenir. La parole est à monsieur Savoldelli pour 10 minutes.

Monsieur le président. Messieurs Ministre, chers collègues. Samedi 3 juin à La Garenne Colombes. Une femme menacée d'expulsion s'est rendu devant la mairie. Ce n'était pas la première fois mais cette fois-ci elle nie demande pas assistance désespérée, elle s'est aspergée des chances en situation de grande précarité. Avec une dette locative élevée et trop peu de ressources pour y faire face à la mis fin à ses jours par l'immolation. Cet exemple dramatique, même s'il n'est pas isolé n'est heureusement pas le lot de toutes les situations de détresse rencontrées par nos concitoyens dans la précarité Séléna commandement de quitter les lieux d'un concours de la force publique et heureusement j'allais le dire. Heureusement parce qu'ils sont 1,2 millions en situation d'impayés. Tout montant confondus. Je prends cet exemple parce qu'il est significatif du désespoir engendré par ces situations de pauvreté et le poids que ce texte peut ajouter sur les épaules déjà bien chargé par les dettes. Véritables criminalisation de la pauvreté. Cette proposition de loi rajoute de la dette à la dette en sanctionnant les impayés par des amendes pouvant aller jusqu'à 7500 euros. Après avoir envisagé d'imposer des peines de prison à celles et ceux dans la misère locative. Plusieurs ici pensent défendent les petits propriétaires. Qui sont de plus en plus minoritaire. En effet, avec 3 5 pour des ménages possédant 50% du parc privé. Il y a des situations d'occupation de logements qui pose problème. Il est vrai, mais elle ne se régleront ni par l'amende ni par la force ni par ce texte. Derrière un texte que vous avez intitulé Loi anti-squats se dissimule des mesures anti-locataire. Le manque de logements accessibles avec des loyers adaptés aux revenus des ménages, le manque de logement tout court, avec un niveau de construction au plus bas depuis 20 ans et bien sûr le manque de places d'hébergement sont des éléments représentatifs du manque de moyens alloués à la politique de logement, avec 5,7 millions de personnes consacrant plus de 35% de leur revenu au logement il paraît évident que seule une revalorisation des salaires et du pouvoir d'achat constituerait une solution pérenne à la crise du logement. Le délai anormalement long pour être reconnus prioritaires au titre du Dalo ne fait qu'augmenter. Il atteint 10 en une décennie, à Paris. Et au moins 3 ans en Île-de-France, et pour beaucoup, partout, les délais sont souvent indéterminé et plus loin encore les hébergements sont toujours saturés insuffisants en nombre comme en qualité. Dans la rue, on ne vit pas, on survit. Si on a de la chance. On est victime de violence, on est confronté à la solitude ou à l'isolement et sans compter la situation des femmes à la rue, victime de l'intersectionnalité de leur situation. Les locataires endettés sont des être s'humains, des femmes, des hommes et même des enfants dans notre pays. Les familles ne sont même pas prioritaire pour un hébergement y compris quand elles ont un enfant si celui-ci à plus de 3 ans. Et là je pense aux jeunes Fallout âgée de 4 ans et à sa maman, passant d'hôtel en hôtel et de logement de secours en logements de secours pendant des mois. Ils étaient livrés à eux-mêmes et dépendant du fonctionnement aléatoire du 115. Sa situation, il y entraîné un retard de croissance inquiétant le jeune Fallout ne grandissait plus depuis ces 3 ans. Hein si mes chers collègues qui vous apprêtez à durcir les sanctions contre les locataires qui se maintiennent à l'abri, sachez que 611 personnes sans domicile sont mortes dans la rue l'an dernier. Et cette année il y en a déjà plus d'une par jour selon le collectif des Morts de la rue, 126 personnes décédées étaient mineurs sur la période de 2012 à 2021 le plus jeune avait un mois en 2021. Cela ne sont-ils pas des enfants comme les autres. La Convention relative aux droits de l'enfant est très clair, dès son article 1er on est enfant jusqu'à 18 ans et dans son article 27 qui demandent le droit à l'alimentation, vêtements et au logement pour tous les enfants. Certains d'entre eux sont des enfants sans toit scolarisés comme le jeune Fallout scolarisés au groupe scolaire de leurs moche à d'Ivry-sur-Seine et je c'est la stupeur des camarades de classe des parents d'élèves, des enseignants face à l'inaction. C'est pourquoi nous avons lutté tous ensemble avec le collectif de parrainage civil de la ville mais aussi et je le reconnais, avec la préfète du Val-de-Marne qui a constaté avec nous l'imperfection des dispositifs d'hébergement d'urgence. Avec la période que nous vivons la hausse des prix dans l'alimentation de l'énergie et tout ça sans avoir de hausse des salaires suffisants, il n'est pas tant de rajouter de la sévérité des punitions allant encon de celles et ceux qui n'y arrive plus pire l'action mises en oeuvre par le gouvernement ces dernières semaines a été de permettent quand même au loyer d'augmenter encore de 3 5 % avec une PPL en séance la semaine dernière PPL que nous avons rejeté mais qui va revenir avec l'aide de la majorité présidentielle de la droite et de l'extrême droite à l'Assemblée nationale. Et comme si tout n'était pas assez cher comme si les appels n'avait pas été les premières cibles de la politique du logement de monsieur Macron dès son premier quinquennat. Le monde vers lequel vous conduisez prend des gens forment il prend forme. 330.000 personnes sont à la rue de 4 millions de ménages attendent un logement social 100.000 dans mon département, le Val-de-Marne, plus de 4 millions de personnes sont mal logées et 12 millions de personnes sont en situation de précarité énergétique. À la bombe sociale provoquée par la crise du logement, vous répondez payé vos loyers où vous paierez des amendes. Pourtant notre droit protège il doit protéger davantage d'abord celles et ceux qui en ont plus besoin, c'est notre rôle d'élu. Notre rôle de républicains convaincus. Alors que les pouvoirs publics n'existe que pour favoriser la cohésion sociale, ils en sont aujourd'hui les destructeurs. Une personne qu'elle soit pauvre ou non. Ah le droit à un toit. Elle a le droit à un logement décent, quelles que soient ses revenus et c'est d'ailleurs le problème de ce texte qui a 100 accentue l'asymétrie de pouvoir entre les locataires et les propriétaires. Avec ce texte vous retirer des droits aux locataires sans ajouter des devoirs aux propriétaires. Comme si le marché règle et tout. J'avais relevé en ce sens les déclarations du président de la République qui, dans un élan de lucidité. Disait il est des biens et des services qui doivent être placés en dehors des lois du marché. C'était le 12 mars 2020 au début de la pandémie de Covid-19 et les promesses du monde d'avant n'ont jamais vu le monde d'après. Les essentiel. Je le cite, que nos sociétés rémunère si mal comme le président de l'ajouter encore compte justement dans le rang, de nombreuses personnes prises à la gorge par le prix exorbitant de leur loyer combinée à la faiblesse de leurs revenus et à la violence de certaines lois. Vous ranger derrière le droit de la propriété. Je viens de l'entendre, c'est là votre seul argument. Alors que ce droit n'est pas mise à mal le propriétaire restant tout à fait propriétaire de son bien qui doit demeurer différentes son domicile là-dessus aussi vous comptez amener plus de flou, avec cette loi en mettant tout sur le même plan la notion de propriété et la notion de domicile. Je le dis avec force le droit de propriété n'est jamais gagnant quand ils s'appuient sur des fondements d'exclusion et d'inégalités d'accès. Et là je veux citer Eugène Varlin, figure de la commune de Paris qui disait très justement. Tant qu'un homme pourra mourir de faim à la porte d'un palais où tout regorgent. Il n'y aura rien de stable dans les institutions humaines. Qu'est devenu le droit au logement, le droit à la dignité et le droit à vivre décemment. Et nous allons déployer notre police et notre justice pour punir les plus pauvres. Je veux vous rappeler les fondements de nos institutions. L'article 2 de la déclaration universelle des droits de l'homme et du Citoyen de 1789, issu de la révolution que nous célébrons avec fierté dans un mois garantit le droit à la vie privée. Cette villa ne peut exister dans la rue. Et comme nous le rappelait l'abbé Pierre. Le logement est un droit et pas un privilège. Les dixième et 11ème alinéa du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 qui ont leur valeur constitutionnelle l'explicite aussi clairement et avec une très grande modernité. Le dixième alinéa, le voici, je vous le site La Nation assure à l'individu à la famille des conditions nécessaires à leur développement. et dit que la nation je cite tout être humain qui en raison de son âge de son état physique ou mental de la situation économique se trouve dans l'incapacité de travailler, a le droit d'obtenir de la collectivité des moyens convenables d'existence. Je vous avoue, je vous pose cette question c'est qu'est-ce qu'on fait ces valeurs constitutives de notre nation. Ne perdons pas de vue l'idéal républicain et ses valeurs qui ont fondé notre république au prix de nombreuses luttes, c'est aussi et j'en termine la demande formulée dans le courrier adressé à la France le 30 mars dernier. Courrier adressé par le rapporteur spécial de l'Organisation des Nations-Unies. Sur le logement convenable et par le rapporteur spécial de l'ONU sur l'extrême pauvreté et les droits de l'homme. Une alerte est aussi formulé. Par l'avis du défenseur des droits. La vie du défenseur des droits, qui trouve ce texte ni nécessaire ni proportionnée. Vous n'êtes pas si sévère avec les marchands de sommeil, l'un d'entre nous l'a évoqué tout à l'heure mais il faut dire les choses. Les marchands de sommeil qui ont une activité lucrative. Et ça vous me direz si je me trompe parce que le garde des Sceaux. Mais il le risque au maximum qu'une amende de 15.000 euros pour profiter de la misère des gens. Donc avec mon groupe nous entendons ces nombreuses alertes unanime et donc nous vous demandons d'acter l'irrecevabilité de cette proposition de loi. Merci pour votre attention. Merci cher collègue. Le président Patriat s'est inscrit pour s'exprimer contre la motion. Il dispose de 10 minutes. Oui j'ai prendrai pas 10 minutes. Monsieur le Président, je prendrai une minute. Sur le président. Messieurs les Ministres, chers collègues, la proposition de loi. Ne porte pas atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution. Elle permet au contraire d'assurer un équilibre entre le droit à la propriété, le droit au respect de la vie privée entre le principe d'inviolabilité du domicile. Et celui du droit au logement. Pour s'en convaincre, il suffit de rappeler que le Conseil constitutionnel le 24 mars dernier a jugé conforme à la Constitution la procédure accélérée d'expulsion qui est prévu à l'article 38 de la loi dite loi Dalo et que la proposition de loi vise à renforcer. Ne Monique ne méconnaît en aucun cas aucun principe constitutionnel. Il est pragmatique et juste. Il aura pour il a pour objectif de rééquilibrer un arsenal juridique jusqu'alors favorable aux occupants. Je rappelle qu'actuellement, mes chers collègues un squatteur risque un an de prison et 15.000 euros d'amende alors que le propriétaire qui change la serrure encourt une peine de 3 ans d'emprisonnement et de 45.000 euros d'amende. Notre objectif n'est pas de mettre plus de difficultés dans la difficulté. Les personnes fragiles mais de trouver des solutions durables pour tous. Il est intolérable de voir se multiplier les sites de promotion de squat. Nous devons être fermes et y mettre un terme. Le squat est entouré d'un mythe politico-romantique qui cadrent qui cache une réalité plus sombre. La détresse de nombreux petits propriétaires souvent sans recours pour toutes ces raisons, le groupe RDPI votera contre cette exception recevabilité. Merci monsieur le président. Monsieur le rapporteur. Monsieur le président, qui a eu l'avis de la commission sur cette motion. Ce le président, mes chers collègues, l'avis de la commission s'André à Pascal Salvodelli et sans surprise défavorable. En première lieu. Parce que l'adoption de cette motion irait à l'encontre de la position exprimée par le Sénat. Déjà en première lecture lors de laquelle nous avons soutenu ce texte qui reprend très largement, je l'ai dit tout à l'heure, les propositions que nous avions déjà voté lors de l'examen de la proposition de loi de Dominique Estrosi Sassone il y a près de 3 ans. Par ailleurs la commission souscrit aux objectifs généraux de ce texte qui nous réussit qui nous réunit aujourd'hui à savoir naturellement la lutte contre le squat d'abord la sécurisation. Des rapports locatifs et la responsabilisation des locataires. Ça a été dit tout à l'heure mais c'est très important que le Sénat substantiellement compléter ce texte en ajoutant un nouveau chapitre renforçant l'accompagnement social des locataires confrontés à des difficultés. Nous pouvons donc considérer ce texte comme plutôt équilibré. Et en second lieu, sur le fond, je souhaite. Répondre aux arguments. Des auteurs de l'exception d'irrecevabilité concernant l'éventuelle inconstitutionnalité du texte non seulement le droit à la propriété privée de longue date, garanti par l'article 17 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Mais le Conseil constitutionnel a également eu l'occasion lors d'une récente QPC rendue en mars dernier de se prononcer sur la procédure d'évacuation forcée qui est amendé par la présente, proposition de loi, le Conseil constitutionnel a alors reconnu que le législateur était légitime, je cite à assurer l'évacuation à bref délai des domiciles illicitement occupé et que ce faisant il a cherché à protéger le principe de l'inviolabilité du domicile le droit au respect de la vie privée et le droit de propriété des occupants réguliers pour ces 2 raisons chère Pascale ça le volet dit. Au titre. Présentant la motion du CRCE. Je vous rappelle, je vous répète que l'avis de la commission est défavorable. Messieurs les ministres qui l'avis du gouvernement sur cette motion. Sans surprise, monsieur le président. Nous avons la même position que celle que vient d'exprimer. Monsieur le rapporteur. Une petite précision cependant puisque vous m'avez invité à l'affaire, si elle était indispensable. Monsieur le sénateur. Savoldelli. Les marchands de sommeil peuvent être punis de 5 ans d'emprisonnement et de 150.000 euros d'amende. Et non pas de 15.000 euros. Comme vous l'avez dit, sans tenir compte d'un certain nombre de circonstances aggravantes. J'ajoute d'ailleurs. Qu'il est parfaitement possible de saisir le dites immeuble. Quand il sert ses hébergements indignes. Et que par des mécanismes que. Nous avons mis en place. On peut aujourd'hui, une fois que l'immeuble et saisis et confisqués cet immeuble peut être réattribué. Notamment à une association caritative. Ce que nous sommes allés faire il y a pas tellement longtemps à Dunkerque. Un dernier mot, et puis je m'assois, monsieur le président, madame la sénatrice Lienemann. La phrase qui vous attend choqué. Je la reprends au mot près. La lutte contre le squat est indispensable. Je pense que vous serez d'accord avec moi et j'ai ajouté. C'est d'ailleurs une de mes priorités. Car oui, la loi doit d'abord protéger les honnêtes gens. Je le confirme. Messieurs. Et ce qu'il y a encore des explications de vote avant que nous nous prononcions sur la motion d'irrecevabilité. une fois deux fois. Je vais donc consulter le Sénat sur cette exception. Je rappelle que l'adoption de cette motion entraînerait le rejet du texte, en discussion. Quels sont ceux qui sont pour la motion d'irrecevabilité. Qui est contre. A été abstentions. Elle est rejetée. Et nous entrons dans la discussion du texte de la commission.

L'amendement numéro 20 sur l'article 1er, Merci monsieur le président. Chers collègues dans ce premier article qui nous est permis de discuter en 2ème lecture. Il reste encore de nombreuses dispositions que nous avions souhaité d'ailleurs retiré en première lecture. Les discussions avaient été intense à l'époque et les arguments. Qui circulaient, qui avait été avancé dans cet hémicycle notamment pour durcir les sanctions contre les locataires en difficulté était en complet décalage avec la réalité du terrain. Les sanctions présentées dans cet article prévoyait même à l'origine des peines de prison contre les locataires en impayés de loyers qui ne quittaient pas leur logement après un jugement d'expulsion. déjà d'une offense à l'égard de nos concitoyens. Quand on connaît la situation de ces familles en détresse et ça a été dit dans les dettes locatives sont souvent pas les seuls menace qui plane sur leur ménage la prison était démesurée. Nous avons obtenu sa suppression et l'amende proposée par est complètement hors-sol, à l'image de ce texte qui généralise des mesures à partir de faits divers en dehors du réel. Il y aurait dans notre pays, des personnes capables de payer 7500 euros d'amende mais qui n'aurait pas été en capacité de payer leur loyer. Alors certes, les loyers sont de plus en plus cher, mais si des personnes n'arrivent pas à payer un deux pièces à 1000 à 1000 euros par mois dans Paris, notamment car c'est la réalité de votre politique du laisser-faire. Croyez-vous qu'ils qu'ils pourront payer les amendes. Certainement pas. Je le redis, notre pays ne manque pas de fermeté à l'égard des locataires les plus pauvres, mais il manque surtout de logements accessibles de places d'hébergement et d'une hausse de salaire qui permettrait à chacun et chacune de payer convenablement son loyer. Merci, chers collègues. Quelle est la ville de la commission sur cet amendement. Monsieur le président. Ce ministre, mes chers collègues, l'avis est défavorable, tout simplement parce que. Cet amendement est contraire à la position du Sénat en première lecture, confirmé par la Commission en seconde lecture. Si Monsieur le Ministre. Même avis monsieur le président. Oui madame. Madame Lienemann souhaite expliquer son vote et de la parole. Je vous l'ai expliqué pourquoi j'étais contre cet article et donc pour la suppression de cet article. C'est qu'il y a une alternative. Il ne faut pas nous faire passer non plus pour des gens qui considèrent que les propriétaires n'ont pas à recevoir le le paiement du loyer et retrouver quand c'est nécessaire. La fin d'un bail, le logement dans un bon état.

D'ailleurs, vous voyez bien à quel point ces risques d'impayés. Temps fort, on est obligé de plus en plus de maîtres des garanties. Je veux même pas parler de l'APL. Or la Gul permettrait à la fois. De garantir le locataire de de bonne foi qui pourraient pas payer le propriétaire toucherait toute de suite son loyer et par ailleurs le le gestionnaire de gueule pourrait se retourner contre les locataires de mauvaise foi, rarement très pauvres d'ailleurs hélas. Et ce système avait été voté par le louer. Or, on ne veut plus parler de ce système de mutualisation du risque à un moment, ils ne font que croître et embellir. Et je vous rappelle, cher Monsieur Patriat que déjà la critique du déséquilibre locataires propriétaires avaient été fait quand la gauche a fait voter en 1981, en l'occurrence 82 la loi Quilliot c'est toujours la même chose, on finit toujours par nous dire que les avancées de la gauche sont pas légitimes ne sont pas bien et du progrès, hélas. Vous faites ah recule sur ce terrain. Je ne vois pas d'autre explications de vote, donc je mets aux voix cet amendement numéro 20 présenté par le groupe communiste, quels sont ceux qui sont pour. Quels sont ceux qui sont contre. Il y a-t-il les abstentions, il n'est pas adopté. Nous avons ensuite 4 amendements en discussion commune dont 2 identique, nous commençons par monsieur Savoldelli l'amendement 22. Oui, merci monsieur le président. Monsieur le Ministre, mes chers collègues. Je ne vais pas vous étonner. Il y a un élément de cohérence entre ce qui a été nos arguments pour les recevabilité. On le retrouve là sur la suppression de l'article de. On pense que c'est une dérive qui était déjà présentes en première lecture. Tout le monde a bien compris hein on va accélérer les procédures pour les expulsions à des locaux qui ne peuvent pas être considérés comme domicile principal d'une personne. Nous, nous considérons qu'il y a pas une urgence a libéré un espace inutilisé ou vacants. Et qu'est-ce qui va se passer on va déployer des forces de police en effectifs, qui sont souvent insuffisants. Dans nos communes. Pour remettre à la rue des personnes. Ces mêmes personnes qui vont se retrouver dans une insécurité. Donc voilà je vous je vous dis ça parce que je ne vais pas développer d'autres aspects du point de vue mais. Je pense que ça sera intéressant dans le débat qu'on a eu et les différentes interventions. On verra quels sont les projets de nos différentes sensibilités politiques quand on abordera le projet de loi de finances. On verra qui encourage à ce qu'il y ait des moyens pour les différents types d'hébergements pour éviter ces situations, merci. En fait cet article permet de pénaliser de 2 ans de prison et 30.000 euros d'amende l'être séduction dans un local à usage David station ou à usage commercial agricole ou professionnel. Pourquoi nous estimant que cette mesure est démesurée régressive et intransigeante.

Nous ne sommes pas opposés à la protection des deux, mais nous souhaitons a minima que la gradation de la protection issu de cette distinction perdure. Autre particularité de cet article c'est la création d'une peine de prison. Nous l'avons vu lors de l'examen de la loi justice la semaine dernière l'inflation pénale crée de fait de plus en plus de comportements illégaux et répréhensible et qui se traduisent de plus en plus. Par criminalisation et pénalisation. Ce qui veut dire incarcération de ces délinquants qui sont très souvent des primo-délinquants. Et ce qui veut dire amplification et l'aggravation du phénomène de surpopulation carcérale d'autant plus que la peine prononcée pour la structure de propriété même inexploité. Montre à quel niveau. Les auteurs du texte pour ce match ce délit par exemple au même niveau que le recel de cadavre. C'est pourquoi nous ne demandons pas la suppression complète de cet article mais de remodeler la peine a fait qu'elle soit ajustés au délit. Un allégement de la peine à un an d'emprisonnement et 15.000 euros d'amende nous paraît déjà plus que largement dissuasif d'autant plus que l'ONU, alerte le gouvernement et rappelle que la France doit respecter ses engagements internationaux et que cette proposition de loi empiète sur certaines libertés les rapporteurs de l'ONU aussi. Nous alertent sur l'extrême pauvreté et les droits humains sur le logement convenable et se penche notamment sur l'Arctique. Nous sommes en train d'étudier en faisant part de leur inquiétude. Nous pensons en ce qui nous concerne que nous devrions réfléchir. Plus l'longtemps sur c'est une sanction qui soit allégée et adaptée. Collègues, ensuite nous avons l'amendement hein rectifier terre le seul signataire dans la salle et Madame Muller-Bronn qui a la parole. Monsieur le président, monsieur le rapporteur. Monsieur le Ministre. L'amendement proposé a pour but de permettre à l'autorité judiciaire de prononcer une interdiction du territoire français. Dans les conditions prévues par l'article 131 30 du code pénal soit à titre définitif, soit pour une durée de 10 ans au plus, à l'encontre de tout étranger qui aurait commis le délit prévu le délit prévu à l'article 315 1 du même code. Le but de la présente loi et de durcir la peine prévue à l'article 315 hein pour lutter contre l'occupation illicite des logements, c'est également le but du présent amendement il convient de rappeler que le respect de la loi pénale et le minimum pour toute personne vivant sur le territoire français aussi. Un étranger qui me méconnaît cette disposition doit pouvoir se voir prononcer une peine d'interdiction du territoire français surtout dès lors que le présent, objet de loi a pour conséquence un durcissement de la peine encourue. Se présente amendement n'a pas pour objet bien sûr de renvoyer tous les étrangers coupables de ce délit. Il a simplement pour conséquence de laisser une marge de manoeuvre plus importante à l'autorité juridique, judiciaire pour prononcer cette peine cette dernière gardienne de la liberté individuelle, conformément à l'article 66 de la Constitution assurera cette nouvelle possibilité dans le seul cadre légal prévu par le code pénal et appréciera chaque situation pour permettre de répondre aux exigences. Demandées par l'état de droit. Merci. De. Monsieur le président, Monsieur le Ministre, mes, mes chers collègues. Cet amendement proposé a pour but de permettre à l'autorité judiciaire. De prononcer. Une interdiction de territoire français que dans les conditions prévues par l'article 131 30 du code pénal soit à titre définitif, soit pour une durée de 10 ans. Au plus à l'compte de tout étranger qui aurait commis un délit prévu à l'article 315 5 du, du même code je crois que c'est le même que celui présenté précédemment et le but de la présente loi et de durcir la peine qui est prévue à l'article précité pour lutter contre l'occupation illicite des logements. Il convient de rappeler que le respect de la loi pénale et le minimum pour toute personne vivant en territoire français aussi. Un étranger qui méconnaît. Ces dispositions doit pouvoir se voir prononcer une peine d'interdiction du territoire français surtout dès lors que le présent. Objet de la loi a pour conséquence un durcissement de la peine encourue. Le présent amendement et ça été rappelé par ma collègue précédemment n'a pas pour but de renvoyer tous les étrangers coupables de ces délits. Il a simplement pour conséquence de laisser une appréciation supérieure une marge de manoeuvre complémentaire à l'autorité judiciaire pour prononcer cette peine cette dernière on le rappelle, est la gardienne de la liberté individuelle, conformément à l'article 66 de la Constitution et assurera cette nouvelle possibilité dans le seul cadre légal prévu par le code pénal et appréciera chaque situation pour permettent de répondre aux exigences demandées. Par l'état de droit. Merci la parole et tout. Rapporteur pour donner un avis de la commission sur ces trois amendements. Sur ces quatre amendements président enfin en plein L'avis de la commission est défavorable sur les quatre amendements. D'une part, au risque de me répéter parce que la rédaction de l'article 1er à nous semblent constituer un point d'équilibre entre les positions exprimées à l'Assemblée nationale et au Sénat et que nous souhaitons qu'ils soient tous adopté conforme. En particulier en entrant dans le détail l'amendement numéro 22 est un amendement de suppression. Il est donc contraire à la position exprimée par le Sénat en première lecture, je le répète. Confirmée par la Commission en deuxième lecture c'est un L4 pardon. Tels qu'ils sont rédigés je m'adresse à. Madame Muller-Bronn. Je m'adresse à Madame, Valérie Boyer tels qu'ils sont rédigés ils autoriseraient le juge a prononcé une interdiction de territoire, définitive pour les personnes étrangères aussi définitif pour les personnes étrangères étrangères condamné pour squat ce qui semble disproportionnée mais. Contraire à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'Homme relatives à la vie privée et familiale. J'ajouterais. Volontiers un argument complémentaire à savoir que. L'article 226 tiré quatre du code pénal qui sanctionne le squat du domicile domicile ne prévoit pas la peine d'interdiction du territoire il apparaîtrait donc disproportionné d'instaurer une peine d'interdiction du territoire pour le squat de locaux à usage économique alors que le squat du domicile bien plus grave en termes de conséquences, on l'a dit tout à l'heure ne le prévoit pas. Sur. L'amendement numéro 9. Les peines encourues pour le squat d'un local à usage d'usage d'habitation ou un squat de local à usage économique ont déjà été abaissée par le Sénat, vous vous en souvenez en première lecture puisque. Le texte transmis par l'Assemblée nationale en première lecture prévoyait une peine de 3 ans de prison et 45.000 euros d'amende pour le squat des locaux à usage d'habitation et de locaux à usage économique soit la même peine que celle que l'article 1er de la proposition de loi prévoit pour le squat de domicile. Nous l'avons abaissé. Nous sommes d'avis à la commission qu'il convient d'en rester à ce compromis qui a été trouvée pour maintenir les fesses dissuasif recherché, je le répète, avis défavorable, c'est le président, mes chers collègues, messieurs les Ministres sur les. Car messieurs rapporteur Monsieur le Ministre, l'avis du gouvernement. Oui, merci monsieur le président, monsieur ça vole des listes d'abord bon comprendrait que je sois totalement hostiles. À l'amendement que vous déposez point n'est besoin. Me semble-t-il d'épiloguer monsieur. Je je je note Monsieur sénateur avec grand intérêt. Que vous n'êtes pas contre le principe de l'emprisonnement. Car vous proposer un an et et 15.000 euros d'amende. Je, je le note avec intérêt. Vous auriez pu proposer un tige. Proposer un an d'emprisonnement. Et enfin le le dernier amendement pardon mais alors si si vous me permettez cette familiarité, on, on y va très très fort parce que si un étranger rentre dans un domicile il ne risque pas d'être expulsés. Mais si il dort sous le hangar. Ils risquent de l'être. Donc au fond votre amendement est incitatif pour l'étranger a squatté le domicile et non pas le hangar qui le jouxte et c'est la raison pour laquelle je suis naturellement totalement défavorable à cet amendement à bien des égards excessif. Madame voyez vous avez souhaité expliquer votre vote. Et C'est pas un caractère définitif, mais je voudrais simplement vous citer un certain nombre de cas. Qui ont beaucoup perturbée nos concitoyens le 10 mai 2022. 104 squatteurs étrangers ont été évacués de 34 logements dans trois bâtiments différents dans la cité Callister à Marseille, le 6 juin 2022. Une personne de nationalité marocaine prétendument mineurs et deux personnes algériennes ont squatté et dégradé une maison à Vienne agressant le propriétaire à son retour, le 26 octobre 2022 à Bègles, 11 personnes algérienne déboutés du droit d'asile sont expulsés d'un squat le 27 janvier 2023 dans le Val de Marne un Tunisien sous obligation de quitter le territoire a été interpellé par la police dans un logement, que des dégradations dont les réparations s'élèverait à plusieurs milliers d'euros. Eu égard à ces différentes situations et il y en a que quelques exemples, malheureusement pas énormément. Concernant les occupations illicites. Il est logique que nous, représentants du peuple français, représentants des communes, nous fassions ce qui est de notre pouvoir pour mieux protéger nos concitoyens, nous ne sommes pas seulement face à des faits divers. Nous sommes face à de véritables faits de société et des drames aussi l'amendement que nous avons proposé a pour but de permettre à l'autorité judiciaire de prononcer une interdiction du territoire français soit définitif, soit pour une durée de 10 ans ou plus à l'encontre de tout étranger qui aurait commis des délits. Du même code contrairement à ce qui m'a été indiqué. l'autorité judiciaire conserve une marge de manoeuvre. Nous ne sommes pas dans une peine automatique ni forcément définitive mais je vous propose une disposition qui reste conforme à l'article 131 troc du code pénal qui prévoit que lorsqu'elle est prévue par la loi la peine d'interdiction du territoire français peut être prononcée à titre définitif ou pour une durée de 10 ans ou plus à l'compte de tout étranger coupable coupable d'un Crime ou d'un délit. Le respect de la loi pénale et le minimum pour toute personne vivant sur le territoire français hein qui méconnaît ces dispositions doit pouvoir se voir prononcer une peine d'interdiction du territoire français surtout dès lors que le présent. Objet

Nous sommes au sénat nous votant des amendements sur des lois, j'ai voté bien entendu l'amendement du groupe CRCE demandant. L'abrogation totale de cet article. Mais il y a aussi bien entendu la possibilité parce que ce que nous votons va concerner des gens de la vraie vie. Des gens qui vont souffrir parce que à un moment donné, voire plus pouvoir payer il va il va falloir qu'il quitte. Les endroits où ça, où ils vont chercher à, à se loger quelque part et ils vont avoir ce délit d'introduction et ces gens-là. Monsieur le ministre, à un moment donné c'est vrai bien sûr que c'est pas l'idéal et bien sûr que je préfère qu'ils soient pas condamnés à des peines de prison. Mais tout naturellement si le juge peut les condamner à 15.000 euros à un an de prison c'était jamais mieux que si peux les condamner à 30.000 euros et 2 ans de prison. Donc ce principe il est exact et ça. Honnêtement je je pense qu'on peut le partager ce qui ne veut pas dire que je souhaite des peines de prison. Je rajouterai une 2ème chose. Et une fois qu'il est condamné, Monsieur le Ministre c'est à nous de faire en sorte qu'il fasse des travaux d'intérêts généraux et qui soit pas incarcéré dans une prison. Parce que finalement à force de condamner des gens et de les mettre dans les prisons, vous aurez beau à construire vous redonner ça suffira pas voilà je parlerais même pas de l'OQTF. Et et des exemples que vous avez cité. Valérie Boyer, parce que des exemples de gens. Qui sont dans des situations dangereuses qui sont dans des situations terribles, voire même qui meurent parce qu'ils ne peuvent pas avoir accès au logement et qui dans ces cas-là, y compris des étrangers vont être obligés d'aller dans des locaux inoccupés pour essayer d'y survivre. Je peux vous en citer autant que ce que vous avez cité comme exemple, y compris à Marseille. Je crois que nous pouvons nous prononcer nous commençons. Le ministre souhaite compléter la discussion. Je serai, je serai taisant dans un instant, je pense que je vais me remettre à l'avis de la commission. Puisque. Nous sommes défavorables à tous les amendements. Mais quand même. je comprends que vous soyez un peu titillés par mon propos qui se veut aimable. Bon à tout pêcheur miséricorde, Monsieur le Sénateur, Madame Boyer. Je vais très très vite. Ce que je disais simplement c'était pas la peine de nous égrener la liste des étrangers qui se sont mal tenus d'ailleurs la liste est assez courte. Je pense qu'il y en a d'autres qui se non, j'ai seulement dit Madame c'est une question de pure logique, vous voyez de pure logique de pure logique. Je dis comment vous portez un amendement. En rappelant que l'étranger qui sont dans un domicile ne risque pas l'expulsion, alors que celui qui irait dormir sous un hangar à la belle étoile risquerait d'être expulsés. C'est tout ce que j'ai dit alors après on peut me faire la liste des Tunisiens, des Marocains, des espagnols qui ont fait six. Ça n'a rien à voir que ce que j'ai dit je suis placé sur un terrain purement logique au fond, vous auriez pu me dire. Que j'avais raison vous n'avez pas souhaité le faire bon moi j'arrête pas polémiquer. Une étude inutilement. Très bien. Donc, nous pouvons voter une que je mets aux voix d'abord l'amendement numéro 22 de monsieur Savoldelli qui a fait l'objet de 2 avis défavorable qui est pour. Qui est contre.

L'introduction d'une amende de 7500 euros en pareille situation est véritablement disproportionnée. Permettez-moi d'ajouter que l'on voit mal comment un propriétaire qui réclame des impayés sera aidé par l'accroissement de la dette de 100 locataire. la réalité ce que cette mesure, le gouvernement n'a qu'un seul objectif, accroître la pression sur les familles et qu'on pourrait leur partout de la même et 8 ans à l'État de trouver lui-même des solutions de relogement avant les expulsions Manu militari. Voilà donc la réponse apportée par la majorité gouvernementale pour répondre à la crise du logement et aux milliers de gens qui éprouvent de gras de difficultés pour se maintenir dans leur chemin. Ce texte il est ni juste ni équilibré. Notre groupe demande que cette sanction pénale soit retiré de ce texte. Entendu. La parole est à monsieur Savoldelli par l'amendement 23 identique. Parfait et ensuite monsieur Ben arrogent défend un amendement 11 qui lui est différent. Merci monsieur le président je je rappellerai juste que monsieur le garde des Sceaux que c'est sur cet article que nous avions fait voter par le Sénat, donc il a été voté ici la suppression de la peine de prison. Voilà c'est juste pour rappeler que je ne suis pas partisan des peines de prison bien d'autres et ça a été conservé par l'Assemblée nationale. Tant mieux.

Parce que nous niveau que le Bastia dans un local désaffecté où dans un local habiter n'a pas la même gravité et qu'une fois de plus la PPL Confo domicile et propriété. Le montant de la de la bande par cet article paraît disproportionné parce que condamner des personnes en grande difficulté financière, à une amende qui va atteindre en fait à peu près 12 fois le montant du RSA. C'est totalement incohérent, y compris pour le propriétaire qui est censé ensuite récupérer de l'argent puisque de toute façon la mode empêchera bien entendu parce que le porte-monnaie de ces gens-là est pas extensible de payer. Ce qu'il doit au propriétaire. Donc ça leur permettra pas de régulariser leur situation, cela aggravera leur précarité et en plus, je rappelle que cette aborde si je ne me trompe pas et cumulative avec la peine déjà très lourde de l'introduction illicite dans un domicile ou une propriété et que le cumul de ces deux peines et suffisamment dissuasif rap dans la bande à 3250 euros pour que nous puissions imaginer justement que le montant de la mode soit réduit si quelques affaires de squat en fait les grands titres et ont permis de légitimer. Auprès de l'opinion publique, la mise en place de cette proposition de loi, la réalité est que cette loi s'attaque aux ménages les plus vulnérables et aura pour conséquence d'empiéter sur leurs droits. Autrement dit, cette loi de ressemblent pas des lots de solidarité de la part des députés Renaissance. Pour être clair. Cet article fait primer la. Il était immobilière sur la nécessité pour elle d'individus de disposer d'un logement je ne rappellerai pas tout ce que dit les rapporteurs de l'ONU à ce sujet juste une phrase qu'il faut donner la priorité voulu aux groupes sociaux vivant dans une condition défavorable en leur accordant une attention particulière. C'est tout ce que nous voulons faire. Monsieur le rapporteur, que ce. Quel est votre avis sur ces trois amendements, dont 2 identique. Alors ces trois amendements reviennent à nouveau sur la position exprimée par le Sénat, lors de la première lecture. Les 2 premiers sont des amendements de suppression. C'est d'autant plus clair. Je voudrais rappeler à cet égard que le dispositif que nous avons voté ne concerne qu'une très faible proportion des locataires défaillants. Il ne s'agit pas du locataire sujet à une difficulté épisodiques de paiement de son loyer mais du locataire défaillant qui se maintiendrait dans le logement en violation d'une décision de justice définitive et exécutoire ayant donné lieu à un commandement régulier de quitter les lieux depuis plus de 2 mois. Concrètement, compte tenu des délais légaux incompressibles qui entoure la procédure judiciaire. Cela signifie que l'on se situer en moyenne déjà 2 ans après le premier. Il semble pour nous non seulement normal mais aussi juste de donner aux propriétaires qui ne peut récupérer son bien un nouvel outil pour dissuader cette pratique. Enfin pour répondre au 3ème amendement donc l'amendement 11, le Sénat, faut-il le rappeler a déjà assoupli le dispositif proposé par l'Assemblée nationale lorsqu'il a supprimé la peine de 6 mois de prison qu'auraient pu encourir ses locataires à baisser en parallèle la sanction pécuniaires risquerait clairement de faire perdre au dispositif toute sa portée. Donc 3 amant 3 avis défavorable. Monsieur le ministre, votre avis. Même avis. Monsieur le Président. Entendu. Donc je mais aux voit s'a des explications de vote. Monsieur Savoldelli vous avez la parole. Merci monsieur le président, c'est non, très très simplement, ce qui, ce qui fait débat. Mais peut-être que c'est utopique. Pour certains, pas juste. C'est ce qui soutient nos amendements que ça soit suppression ou des fois des amendements de repli. Fait par la gauche. C'est de partir du principe que quand on s'opère nos on exécute une expulsion. Il y a une alternative de logement. D'hébergement même voilà c'est cette question là qui fait débat. Je suis pas sûr qu'elles appartiennent qu'à la gauche. Mais ça c'est une vraie question. Parce que quand on exclut quelqu'un ou une famille. Elle se retrouve à la rue et je pense que. C'est pour ça que je vous disais tout à l'heure les valeurs républicaines. C'est pas de proposer. N'importe quel hébergement à n'importe quel prix et caetera bêtes proposées au moins un hébergement.

c'est de penser que quand on en arrive à à cette étape là, on est en devoir. La République de faire une offre d'hébergement. Là c'est pour qu'on comprenne bien la la nature de nos amendements. Je vous en remercie. Je ne vois pas d'autres demandes d'explications de vote, donc je mets aux voix l'amendement six de monsieur Bois-d'avec 2 avis défavorable qui est pour. Qui est contre. Il y a pas d'abstention il est pas adopté. Et c'est même vote sur l'amendement 23 forcément parce il est identique. Et sur l'amendement 11 monsieur Bena Roche avec également 2 avis défavorable qui est pour cet amendement. Qui est contre. Y a-t-il des abstentions il n'est pas adopté et nous pouvons donc nous prononcer sur l'artistique. Le 1er a donc non modifié. Qui est pour l'article 1er, Qui est contre l'article. Est-t-il des abstentions il est adopté. Le 1er essai est maintenu en suppression donc sa suppression est maintenue, pourrait français. Sur la l'article de nous en sommes à l'amendement 26 de monsieur Savoldelli qui ouvre la discussion. Il est défendu que de l'avis de la commission sur cet amendement de suppression. Défavorable car contraire à la position du Sénat en première lecture. Monsieur le Ministre défavorable. Explications de vote, je n'en vois pas, donc qui est favorable à cet amendement 26 de monsieur Savoldelli. Qui est contre. Y a-t-il des abstentions il n'est pas adopté. Nous avons ensuite trois amendements en discussion commune.

les des alinéas précis dans cet article que nous aurions souhaité voir disparaître et qui étend les procédures d'expulsion accélérée en mettant sur le même plan tout type de propriété vous ne protégeaient pas seulement les logements contre l'occupation illicite mais vous empêcher toute mise à l'abri de quiconque, quelles qu'en soient les raisons ou quel que soit le lieu d'ailleurs il est un fait. Que vous êtes en train de franchir une nouvelle étape pour durcir encore les mesures à l'encontre des plus précaires en renforçant la protection des biens au détriment des des personnes. Alors c'est vrai que respecter la propriété s'ans mais expulser sans solution de relogement de relogement et c'est ce que vient d'évoquer, mon collègue ou de mise à l'abri, ce n'est pas défendre l'intérêt général. L'espérance de vie dans la rue, nous le savons, elle est d'environ 50 ans et pour celles et ceux qui s'en sortent et qu'qui quitte la rue c'est souvent avec des séquelles et de grandes difficultés de réinsertion qui forment un cercle vicieux que ce texte va inéluctablement compliquer davantage. Alors d'une part il faut. Éviter les expulsions à tour de bras et puis je voudrais apporter une petite précision. J'avais constaté à la fin de l'année 2022 2000 enfants nuit à la rue. Chaque nuit, ils sont sans toit ni loi pour les protéger. C'est une situation que je considère pour ma part insoutenable. Elle est indigne de notre pays signataires de la convention internationale des droits de l'enfant. Ensuite l'amendement 13 monsieur Bena Roche. Cette présente, proposition de loi en fait ouvre un nouveau paradigme très clairement. Ma collègue vient de le dire avec d'autres mots ce paradis mais il est porteur d'une grande violence sociale, c'est le paradis de la primauté absolue du droit de propriété sur toute autre droit social et notamment sur le droit de disposer d'un logement pour vivre. Le Conseil constitutionnel. Pourtant, en 1995 déjà avait érigé la possibilité pour toute personne de disposer d'un logement décent au rang d'objectif de valeur constitutionnelle. cet amendement, nous en sommes les auteurs parce que nous souhaitons dénoncer en particulier donc la dénaturation insidieuse du délit de violation de domicile et de la procédure d'expulsion prévue en conséquence. Pensé pour protéger la vie privée des personnes en sanctionnant l'occupation de logements meublés et régulièrement habiter le délit protège désormais la propriété immobilière en sanctionnant l'occupation de tout local d'habitation futile inhabité vide de tout meuble ou vacants depuis des années. Cette extension considérable du délit de violation de logement et d'autant plus chocottes. Monsieur le Ministre du logement que la France compte aujourd'hui 10 fois plus de logements vacants que de personnes à la rue.

l'amendement numéro 136 qui avait été déposée en novembre 2022 a été adopté en première lecture à l'Assemblée nationale et il prévoit bien d'élargir la faculté de constater l'occupation illicite constitutive d'un squat de domicile. Au maire. En effet, ils rappellent que le maire exerce d'ores et déjà ses attributions d'officiers de police judiciaire sous la direction du procureur de la République. Il s'agit d'une avancée importante, même si le présent présent amendement propose de rajouter également la possibilité pour les adjoints de procéder à ce constat pour rester en cohérence avec le premier alinéa de l'article 16 du code de procédure pénale. L'amendement numéro 136 rappeler également que comme les auditions, l'ont montré les officiers de police judiciaire sont bien souvent insuffisamment nombreux pour pouvoir procéder au constat de manière réactive. En effet le renfort du maire ou de ses adjoints dans cette procédure ne sera pas inutile mais restera insuffisant notamment dans certaines communes de grande taille ou de taille moyenne. Le présent présent amendement a donc pour objet de permettre également aux agents de police judiciaire de procéder à ce constat. Les agents de police judiciaire sont sous les ordres et sous la responsabilité des officiers de police judiciaire. Ils ont pour mission de constater les crimes, délits et contraventions et d'en dresser procès-verbal. Ils sont donc tout désigné pour pouvoir également procéder à ces constats donc une extension pour les adjoints au maire et pour les officiers de police judiciaire. Merci. Exactement monsieur le président. Je vous remercie, c'était exactement le même. C'est la raison pour laquelle. Je ne vais pas revenir sur l'exposé des motifs mais. Répondre par anticipation à aux échanges que nous avons pu avoir en commission parce que vous le savez, il était prévu jusqu'à présent à l'article 38 de la loi du 5 mars 2007. Je cite, qu'en cas d'introduction et de maintien dans le domicile d'autrui qu'il s'agisse ou non de sa résidence principale à l'aide de manoeuvres, menaces voies de fait ou de contrainte, la personne dont le domicile est ainsi occupé ou toute personne agissant dans l'intérêt pour le compte de celle-ci peut demander au préfet de mettre en demeure l'occupant de quitter les lieux après avoir déposé plainte fait la preuve que le logement constitue son domicile et fait constater l'occupation illicite par un officier de police judiciaire. Les députés ont élargi cela aux maire et aux commissaire de police. En effet, comme les auditions leur montrer à l'Assemblée nationale. Les officiers de police judiciaire sont bien souvent insuffisamment nombreux pour pouvoir procéder au constat de maintenir réactive en aucun cas il n'a été prévu que les adjoints au maire et les agents de police judiciaire puisse avoir cette faculté de constater l'occupation illicite constitutif d'un squat de domicile. Si le Parlement a été capable d'élargit sa faculté aux maires et au commissaire de police pourquoi ne pourrions-nous pas le faire pour les agents de police judiciaire où les adjoints au maire. Si cela n'était pas prévu pour les mères ou les commissaires pourquoi il serait prévu pour les agents de police où les adjoints au maire. amendement le même amendement que que ma collègue Madame Muller-Bronn n'a qu'un seul but c'est accélérer le déroulement de cette procédure afin d'expulser les squatteurs au plus vite et c'est aussi faire en sorte que les mairies soit plus efficace et soit moins soumises. Aux aléas de ses occupations pour chacun d'entre nous a pu le constater quand on a été maire, hé bien nous avons souvent affaire à des victimes de squat et on ne peut que mettre en place des procédures qui sont longs, qui sont lourdes, elles sont améliorées mais celle-ci permettrait d'être beaucoup plus réactif, je vous remercie. Merci monsieur le président. En fait notre groupe trouve disproportionnée la possibilité d'utilisation. Du régime d'exception de l'article 38 de la loi Dalo lorsqu'il s'agit de locaux vides. Dans les locaux vides, quoi faire. Monsieur le. Garde des Sceaux. Polnareff disait dans la chambre vite, je passe mon temps à regarder dans la maison vide, moi je vous dis monsieur le garde des Sceaux, est-ce qu'on peut utiliser une une une exception de, d'utilisation de la loi Dalo lorsqu'il s'agit de locaux vides. vides. Les délais d'évaluation plus la situation personnelle sur tellement court et la non-judiciarisation de la mise en demeure. Dans ces cas-là. Ne nous paraît pas justifié. Je rajouterais juste une chose puisqu'il me reste une minute. Quel ça m'évitera d'en parler après. Il y a un autre amendement. Auquel nous tenions particulièrement ça a été évoqué tout à l'heure dans une déclaration générale ou dans la motion des recevabilité.

je ne sais pas pour quelle raison cet. Amendement-là a été jugé comme entrant dans un entonnoir dont il n'est donc jamais sorti. Pourtant, les marchands de sommeil je ne vois pas quel est leur tout noir en l'occurrence mais bon et puis les marchands de sommeil. Pour autant, c'est quand même un vrai problème. L'avis de la commission. Monsieur le rapporteur. Sur ces cinq amendements dont 2 identique. L'avis de la commission sera défavorable sur ces cinq amendements. S'agissant des amendements de suppression donc 24 et très ils reviennent explicitement sur la position exprimée par le Sénat en première lecture, je considère que. Nous avons par conséquent déjà largement plus débat de ces sujets.

afin de prendre en compte les récentes réserves d'interprétation, que le Conseil constitutionnel a formulé à l'occasion d'une QPC. J'en ai parlé tout à l'heure ces ajouts de l'avis de la commission sont utiles et garantissent la pleine conformité de la procédure d'évacuation forcée de l'article 38 de la loi Dalo à la constitution. Il est donc souhaitable de maintenir ce grand trois. En outre ces amendements je regarde particulièrement. Valérie Boyer sont partiellement satisfait puisque les adjoints au maire, tout comme les maires ont déjà la CAF qualité d'officier de police judiciaire, conformément à l'article 16 du code de procédure pénale et à ce titre, ils peuvent donc déjà constater l'occupation illicite d'un logement. Enfin concernant l'amendement 10 monsieur Bena Roche. Il me semble aller à l'encontre de son objet. Sûrement aux dépens de ses auteurs puisque le dispositif de cet amendement vise à supprimer les alinéas qui permettent de différer l'expulsion. Qui permettent de différer l'expulsion je vous invite donc. Vous et vos collègues de du groupe gestes à le retirer. Parce qu'effectivement je pense qu'il va vraiment pas dans votre sens, ou à défaut l'avis sera défavorable, je vous remercie. Elle avait ensuite du gouvernement, Monsieur le Ministre. C'est 5 fois le même avis défavorable, monsieur le président. Madame Lienemann a souhaité expliquer son vote là. Oui, moi je voudrais soutenir les amendements, notamment notre collègue Bennaoum. Concernant la la différenciation entre l'occupation d'un domicile et d'un autre local. C'est vous, vous êtes en train de rompre un équilibre entre l'intérêt général, l'ordre public et la propriété qui a été finalement défini à partir de la Libération. Le vrai CNR. Monsieur le Ministre. Puisque il avait été considéré à l'époque. Que l'intérêt général et l'ordre public. Justifiait notamment la réquisition de logements ou de Dabou de locaux vides. Au motif que la propriété pouvaient être entre guillemets interrompu dans un dans son un usage au motif de l'intérêt général de l'Ordre public et du droit au logement, la dignité des personnes. Et là pour le coup, ce droit de réquisition était totalement impossible s'agissant d'un domicile. D'une famille. Ces débats. Ils ont lieu depuis cette période là. Quel est le bon équilibre entre le droit de propriété. L Usu ça bug ZUS c'est-à-dire. Abusé de sa propriété. Pour ne rien en faire. C'est un vieux débat. et là vous rompez complètement cet équilibre qui avait été trouvé de plus d'un. Dès cette époque sur ces 2 conceptions, je crois que c'est un gros recul républicain. J'espère que l'histoire. Montrera qu'il vaut mieux revenir aux législations antérieures. Je ne vois pas d'autres explications. Oui Madame Boyer pardon je l'avais vu et j'allais oublier. Monsieur le rapporteur. Chers collègues. Je je vais retirer mon amendement parce que. Vous vous m'avez satisfait avec Response. La difficulté est la raison pour laquelle nous avons développé déposé cet amendement pardon c'est parce que. Il est peut être satisfait. Juridiquement, mais il ne, il n'est pas effectif. Donc j'espère qu'à l'issue du texte, quand tu nous l'aurons voté.

voilà parce que pour l'instant on s'est renseigné et si on a déposé cet amendement, c'est parce que ça ne fonctionne pas sur les territoires et qu'aujourd'hui on a vraiment besoin de ces dispositions. Je vous remercie. Merci cher collègue. Alors il ne reste donc l'amendement 24 de monsieur Savoldelli d'abord avec double avis défavorable qui est pour.

Contre. Ça. L'abstention est pas adopté ensuite toujours sur l'article de. Il nous reste un amendement qui le 21 monsieur Savoldelli qui le présente. Oui, merci Monsieur le Président, messieurs les ministres, mes chers collègues. Je l'évoquais tout à l'heure, qu'est-ce que pose cet amendement, c'est qu'il n'y ait pas d'évacuation forcée qui soit réalisé quand il y a aucune place d'hébergement qui peut être proposer aux occupants du lieu. On a tous notre parcours et notamment moi je connais un peu pas intimement mais un peu le partout. Cours du ministre du Logement. Donc il il sait et il connaît ces situations-là, moi je l'ai connu dans mon département avec l'action sociale. On le sait. Les travailleurs sociaux, ils appellent ça le fonctionnement en l'escalier. Je crois que ça vous parle. Les travailleurs sociaux, parce que quand vous vous entrez dans un hébergement d'urgence. Vous devez ensuite obtenir avec un hébergement de réinsertion sociale avant d'avoir un droit au logement de droit commun. Je, je vous dis ça parce que. Franchement. Il faut, il faut qu'on arrive à trouver quand même une réponse à ça. Quand on voit que les chiffres ont explosé. On dit 330.000 mais c'est un recensement d'ailleurs que d'aucuns conteste ici Mais je pense qu'on est au dessus même. Mais si on continue à ne pas trouver. Des réponses d'hébergement. On va aller à une situation d'une violence extraordinaire dans notre société

Donc moi j'attire votre attention là-dessus, c'est le sens de de cet amendement. Et vous pourriez demander aux travailleurs sociaux les difficultés qu'ils rencontrent et là c'est pas une dimension idéologique c'est que ils ils vivent cette situation l'escalier.

Monsieur le président. Monsieur le Ministre, mes chers collègues. Moi je voudrais vraiment dire à Pascal. Savoldelli je suis sensible à son argumentation qu'il qu'il réitère à l'instant. Mais je voudrais vraiment attirer son attention sur le fait que d'ores et déjà le préfet dispose d'une marge. D'appréciation, avant de décider de mettre en demeure un squatteur de quitter le domicile d'autrui dans sa rédaction actuelle de l'article 38 de la loi Dalo autorise le préfère ne pas donner suite à la demande d'un propriétaire victime d'occupation frauduleuse son logement s'il estime qu'il existe, je cite, un motif impérieux d'intérêt général comme vous le savez les marges d'appréciation du préfet ont même été accrue lors de l'examen du texte en 2ème. Lecture à l'Assemblée nationale pour tenir compte de la récente QPC j'en ai parlé tout à l'heure, il est désormais prévu que le préfet. Considère je lis la situation personnelle et familiale le l'occupant. L'occupant illicite si s'il en est. Avant de prononcer une mise en demeure. Ces précautions. Me paraissent satisfaisantes sauf à à nier. La possibilité d'intervention. Du du préfet. Elle me paraissent proportionnées afin de maintenir l'effectivité du dispositif qui s'adresse, je le rappelle aux squatteurs de domicile d'autrui et non aux locataires défaillants, qu'on en soit hein, c'est encore mieux de le rappeler une nouvelle fois. Donc malheureusement, je répète, je comprends tout à fait. La sensibilité du groupe CRCE à l'égard de de ce de ce, de ces problématiques. Mais pour les raisons indiquées, je donne un avis défavorable. Et l'avis du gouvernement féministe. Je ne vois pas d'explication de vote si j'envoie une monsieur Savoldelli qui a la parole. Tout à l'heure, le garde des Sceaux ma sûrement repris sur les amendements, les amendes concernant et les sanctions, y compris pénales par rapport aux marchands de sommeil. J'aurai intérêt pendant la diligence du moment mais je serais intéressé vous me fassiez parvenir les les dernières décisions qu'il a eu concernant les marchands de sommeil. Ça m'intéresse parce que si je me suis trompé, je reconnais mes erreurs et de j'ai j'aime bien me conformer à à la à la vérité, donc je suis intéressé que vous me donniez les éléments sur les décisions de justice concernant les, les marchands de sommeil. Par contre je vais, je vais vous dire une chose. Mes chers collègues, c'est si j'avais dit tant d'énormités. Tous repris j'en doute pas, j'ai l'habitude ici d'un débat aiguisé argumenté. Mais à Paris, c'est 10 ans le Dalo. 10 ans en moyenne. 3 ans en Île-de-France. Donc je j'en, j'entends l'argument sur le préfet va prendre, prendre des mesures et après mais il faut, faut voir ce qui se passe. c'est pas le préfet qui est en cause c'est pas la clé où la préfète. C'est que ça c'est factuel. Mes chers collègues. C'est 10 ans à Paris, 3 en Île-de-France. Et et dans vos départements vos régions de ce que j'ai j'ai quand même des collègues qui ne sont pas d'Île-de-France. Les délais ne cesse d'être de plus en plus long. Donc je vous dis ça voilà. Ça c'est factuel. Donc j'attire notre attention collective. Sans polémique. Mais on va aller à une extension hein non quantitatif. Exponentielle de gens qui vont se retrouver sans toit, sans hébergement. Si on ne trouve pas une alternative. Vous vont passer au vote sur cet amendement numéro 21 qui fait l'objet de 2 avis défavorable qui est pour. Qui est contre. Il s'abstient. Il n'est pas adopté. Nous en venons au vote sur l'article 2 également inchangé. Qui est pour l'article 2.

Sur cet amendement, le texte pérennise un dispositif qui autorise les propriétaires a confié la gestion de leurs biens immobiliers vaccin à des sociétés privées, agréées par l'État. Qui passe dans des lieux des résidences des résidents temporaires du Rhin une période limitée en échange d'une redevance des lois successives en prévu que ce dispositif aspirine mental devait faire l'objet d'une évaluation remise au Parlement. Aucun rapport n'a été remis ou transmis par le gouvernement. Par ailleurs, il semble que ce dispositif soit justement perfectible, compte tenu des remontées de terrain dans ton disposons. Il est pour le moins surprenant de pérenniser un dispositif alors même que plusieurs médias ont récemment dénoncé dénoncer des dérives qui mériterait au contraire de revoir les conditions de délivrance et de contrôle de l'agrément de l'État ainsi que les conditions sanitaires et le respect de la vie privée sans évaluation de la part du gouvernement. Notre groupe sera opposé à Périnne pérennisation de ce dispositif. Monsieur ben rôle vous bien défendu un amendement identique le 17. On a souvent critiqué cette façon d'avancer ici pour toute tata d'expérimentation qui a été menée et nous tout ça sur tous les bancs quelques quelques quelques quelques groupes que nous soyons là en fait je rappelle juste un truc quand même si ça a été mis en place, expérimentation en 2009. Il devait y avoir un rapport annuel du de suivi et d'évaluation chaque année de 2010 à 2014, 5 rapports. La loi Alur de 2014, elle a prévu la communication au Parlement d'un rapport biannuel de suivi et d'expérimentation de fin 2015 à 2018, 7 rapports. La loi an 2018 à proroger l'expérimentation rappelant l'obligation de fournir un bilan avant le terme de l'expérimentation au 31 décembre 2023, soit un rapport que qu'on a toujours pas vu. Donc au total ça fait 13, rapport qui ont pas été remis. Et là où nous demande de généraliser une expérimentation qui n'a jamais été évaluée dont aucun rapport d'évaluation a été remis 13 rapport par des gouvernements successifs. Je, je ne comprends pas la cohérence de d'autres céda aujourd'hui avec tout ce que nous avons voté par le passé pour transformer. Cette expérimentation généralisation sur la remise d'aucun rapport depuis 2009.

à l'occupation temporaire que la loi Elan lui a pourtant confié explicitement. Il serait cependant malvenu de refuser la pérennisation d'un dispositif pour la seule raison de l'inaction du gouvernement, je le dis comme je le pense. La pérennisation permettra au contraire d'apporter une sécurité juridique aux propriétaires qui mettent à disposition leurs locaux, ce qui leur permettra les auditions que j'ai d'ailleurs pu mener en qualité de rapporteur ont permis de dresser un avis favorable de cette expérimentation, selon les chiffres qui m'ont été transmis plus de certes avant la première lecture. Plus de 1000 bâtiments vacants ont fait l'objet d'une occupation temporaire depuis la création de ce dispositif, ce qui a permis de loger près de 10.000 résidents temporaires. Ces chiffres démontrent que ce dispositif a trouvé son public et mériterait d'être davantage connu aussi bien pour lutter contre la vacance des logements que pour proposer des solutions d'hébergement temporaire. Enfin, je voudrais rappeler que l'Assemblée nationale a adopté un amendement qui impose à l'État de procéder à des contrôles réguliers des associations et organismes qui bénéficient de ce dispositif. Dans ces conditions, il nous semble opportun de pérenniser ce dispositif qui a d'ailleurs été, faut-il le rappeler prorogé déjà à 3 reprises. C'est pourquoi j'aimais un avis défavorable à ces amendements. Quel est l'avis du gouvernement, Monsieur le Ministre. Merci monsieur le président. J'ai j'ai mettrait aussi un avis défavorable et et je maintiens le le souhait du gouvernement de de pérenniser. Ce dispositif, le vieux prof de sciences physiques que je suis à tendance avancée qu'une expérimentation de de 14 ans n'est plus est tout sauf une expérimentation mais une pérennisation déguisé effectivement les les l'évaluation. N'a pas été faite par plusieurs gouvernements depuis 14 ans et je le regrette mais nous allons à mettre en place une mission d'inspection pour que ce dispositif qui pour l'essentiel fonctionne bien soit pérennisé si des organismes. Devaient être défaillance qui a parfois été le cas, hé bien je me suis déjà engagé, nous leur retireront leur agrément mais en attendant je pense qu'il, il faut être défavorable ou un retrait à cet amendement. Merci. Je vais mettre aux voix, ces deux amendements identiques, les 8 et 17. Sauf si quelqu'un demande, a expliqué son vote. Qui est pour ces amendements avec double avis défavorable. Les 8 et 17 de monsieur madame

j'espère juste que les contrôles qui sont prévus du gouvernement se déroulera au réellement et qu'on aura effectivement des informations. Sur les contrôles, puisqu'on n'a pas eu des informations sur l'expérimentation. Cela étant dit, Monsieur le Ministre, je pense que c'est bien qu'il y a des contrôles. Cela étant dit on pourrait à défaut. Au moins essayer d'encadrer un petit peu puisqu'on en sait très bien qu'il a des dérives hein. Tout se passe pas forcément aussi bien dans le meilleur des modes même si ça se passe bien. Certaines fois ça se passe mal d'autrefois, vous le savez très bien donc. Parmi les mesures possibles d'encadrement on en propose une, Qui est celui. De renforcer les conditions de délivrance et de contrôle de l'agrément de l'État. Pour les opérations d'occupation temporaire des locaux. En limitant leur compétence territoriale c'est-à-dire lieu là d'accorder à d'agrément ouvert partout à des sociétés qui sont souvent des sociétés de gardiennage. Je pense qu'on pourrait mieux les contrôler. Si on commençait par limiter les les autorisations ou les agréments. À certains territoires donc avec une compétence territoriale. Entendu quelles sont qu'est l'avis de la commission sur cet amendement de monsieur le rapporteur. Le 15. C'est un, un avis défavorable dans la mesure où il est déjà satisfait l'article 1er du décret d'application de l'article 29 de la loi Elan qui régit ce dispositif d'occupation temporaire de local vacant prévoit explicitement que la demande de l'agrément et présenté par l'organisme ou l'association intéressé au préfet du département où si situe une des opérations d'occupation temporaire envisagée donc. Avis. Proposition de retrait. Sinon, avis défavorable. Ensuite. L'avis du gouvernement. Même avis. Monsieur le Président défavorable. Vous le maintenez, monsieur blanc rouge. Je mets aux voix l'amendement 15 de monsieur. Avec double avis défavorable qui est pour cet amendement. Qui est contre. Il y a pas l'abstention est rejeté. Nous passons à l'amendement 27 de monsieur Savoldelli. Oui alors là il s'agit. On a aussi des. Une demande d'évaluation. Mais puisque le dispositif est maintenu, nous préconisons qu'. Une personne puisque normalement le bas il s'arrête parce que l'opération d'aménagement ou parce que le, les travaux dans le le bâtiment doivent se mettre en oeuvre et nous considérons qu'à partir du moment où les travaux et l'aménagement n'aurait pas lieu. Puisque normalement c'est doit avoir lieu de trois mois après le départ de la personne. La personne qui resterait dans les lieux en payant évidemment le loyer ne pourrait pas être expulsés tant qu'évidemment il y a pas les signes tangibles du démarrage des travaux de l'aménagement. Et la ville de la commission. Monsieur le rapporteur. La proposition de nos collègues du groupe CRCE aurait simplement pour effet de dissuader de nombreux propriétaires de locaux vacants de les mettre à disposition pour une occupation temporaire. la période de vacances est supérieure à trois mois par exemple. Le temps pour le propriétaire de trouver les fonds nécessaires à la réalisation des travaux d'ampleur les dispositions relatives à la libération des lieux par les occupants temporaires ne seraient plus applicable l'instauration d'un régime différent selon que la vacance supérieur ou inférieur à 3 mois rendrait en outre à mon sens le dispositif moins lisible plus complexe, je le répète un effet induit de cet amendement serait que. Le dispositif de l'article 29 de la loi Elan. Ne trouverait plus de de de de de propriétaires intéressés. Donc, avis défavorable du gouvernement, monsieur le ministre. Mot pour mot le même avis que le rapporteur défavorable. Je mets aux voix cet amendement 27 avec double avis défavorable qui est pour. Qui est contre. Ah l'abstention il est adopté, il y a le 28 ensuite qui est présenté par Monsieur Savoldelli. Oui, merci monsieur le président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues. Cet amendement propose une mesure relativement modérée. Qui s'apparente d'ailleurs aux dispositions réquisitions qui ne sont jamais employé par les préfets là-dessus, je ne sais pas si Madame Valérie Boyer va nous faire une liste complète des réquisitions par les préfets. Ça va être difficile à mon avis. Pourtant ils ont le droit dans la loi. En ce qui concerne les logements vacants. Avec l'alinéa. Nous proposons d'ajouter il y aurait la possibilité pour le préfet ou la préfète de prolonger une occupation éphémère en renouvelant le contrat de résidence temporaire et ainsi conserver la protection existantes à l'égard d'une personne sans domicile. Donc cette nouvelle disposition pourrait notamment avoir une utilité. Bon je pense particulièrement et tout le monde le sait ici, quand il y a des périodes de grand froid. Quand on a on a des difficultés, c'est le moins qu'on puisse dire, à avoir des places d'hébergement suffisantes ou des personnes s'apprêtent à se retrouver dehors et augmenter les effectifs des personnes sans domicile fixe. Voilà, nous vous proposons là, c'est une mesure concrète, c'est une alternative qui permet aux préfère. D'autoriser une occupation éphémère temporaire sous le contrôle de l'État. Donc là si on dit non aussi à cette proposition. Je m'excuse, la dette un peu. Directif peut être clivant pour certaines et certains mais ça veut dire que vraiment on cherche pas à trouver une solution à quelqu'un et donc on le renvoie à ne pas avoir un toit et ne pas être hébergés. Et de l'avis de la commission. Monsieur le rapporteur, sur l'amendement 28. Je ne suis vraiment désolé pour pour Pascal Salvodelli. Mais comme pour l'amendement précédent la position de nos collègues du groupe CRCE aurait pour effet de dissuader de nombreux propriétaires de locaux vacants de la mettre à disposition pour une occupation temporaire. Ce dispositif assurément ne peut fonctionner que s'il reste suffisamment souple, aussi bien pour le propriétaire des locaux que pour les résidents. En outre. Parce que j'ai essayé de voir dans quelle mesure, compte tenu de la sensibilité qui est la vôtre. Cher collègue à à cette nécessité de de de solutions alternatives d'hébergement. Telle qu'il est rédigé cet amendement permettrait à des résidents temporaires de se maintenir dans le logement indéfiniment puisque. La période de 6 mois mentionnés par l'amendement serait renouvelable. Et donc l'avis de la commission est défavorable. L'avis du gouvernement, Monsieur le Ministre. Même avis monsieur le président. Madame Lienemann et monsieur Savoldelli explique chacun leur vote. Oui. J'ai bien compris monsieur le rapporteur. Votre thèse que à la limite je peux encore entendre. S'agissant d'un droit qui serait donnée à une personne. Un peu automatiquement. Si le, l'opération n'a pas lieu. Là il s'agit de donner aux préfets. La possibilité de juger de l'opportunité. Et vous savez très bien que le préfet va pas s'amuser. À faire quelque chose qui serait de nature à empêcher une un prochaine aménagement de la construction et par plus plaisir nuire à un propriétaire qui aura un projet. Donc le fait que ce soit le procès le préfet qui décide permet justement de juger du bon équilibre entre la réalité du projet l'intérêt et de maintenir cette personne parce que vous savez aussi il y a des gens qui pensent qu'ils vont pouvoir faire leurs projets dans 3 mois 6 mois puis qui savent qu'il y a retour il y a un retard pour X raison. Des permis de construire, contesté, des choses comme ça qui fait que, avec même avec le préfet. Un accord peut être trouvé. C'est pourquoi nous pensons que dans le cas où il s'agit d'autoriser le préfet à prolonger ce bail temporaire. On n'est pas du tout dans un cas aussi dissuasif que vous pouvez. Le craindre. monsieur le président. Je vais être très court mais Marie-Noëlle Lienemann a bien explicité la nature, alors il y avait aucune mauvaise volonté du froid porteur. Mais là c'est pas le droit de la personne. C'est sous l'autorité des préfets. Avec une proximité de reconduction au bout de six mois. Enfin franchement. Ayons confiance dans les représentants de l'État. Dans le département. je ne vois pas où est le doute là enfin je veux dire voilà. Donc je pense que je, voilà ce que je vous demande c'est. Vous allez voter ce que vous voulez mais il faut voter par rapport à la réalité de cet amendement. Cet amendement autorise donc une occupation temporaire. Éphémère. À l'initiative et par un diagnostic du préfet. Donc c'est ça qu'il faut voter oui ou non les préfets pas avoir cette condition de souplesse par rapport à une situation donnée. Monsieur Benalla Roche. Oui j'apprécie toujours des arguments de monsieur le rapporteur. Parce que effectivement. Il défend le fait que le texte ne va pas bouger, il défend chaque amendement et je l'remercie. Là ce que je ne comprends pas en fait d'une manière ou Montety qu'on peut considérer que l'argument. Monsieur le rapporteur, consisterait à dire en fait le propriétaire fait pas confiance à l'État. pas à celui qui occupe mais le propriétaire fait pas confiance à l'État pour faire respecter le droit de propriété. C'est ça en fait que ça veut dire. Enfin s'il fait pas confiance à l'État et peu au fait au moins faire confiance au Sénat parce que ça je sais qu'au Sénat, le droit de propriété. Vous allez le défendre. Donc en fait il y a pas de risque pour le propriétaire monsieur le rapporteur. Nous pouvons passer au vote sur cet amendement 28 avec toujours de l'avis défavorable qui est pour. Qui est contre. Il n'y a pas d'abstention il n'est pas adopté, nous pouvons voter sur l'article de terre également inchangé qui est pour l'article de Qui est contre. Il est donc adopté. Nous avons quelques amendements sur l'article IV. Et nous commençons par un amendement 29 de monsieur Savoldelli. Oui, merci Monsieur. Le président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues. Il s'agit de l'article 4. Dans le. Et. Sans prendre de raccourci. Qu'est ce que propose cet article 7 systématiser la présence de clause de résiliation dans les contrats de bail. Moi, je nous nous pensons notre groupe. Mais c'est aussi le fait de d'associations. Et de, de beaucoup de nos concitoyens. Qu'on ne peut pas. Penser un seul moment que toutes les situations sont identiques. Et ça a été dit tout à l'heure d'ailleurs tous les impayés sont se justifie pas par une expulsion. Et qu'un contrat de location s'appuie sur d'autres piliers qu'une simple question de paiement. j'attire l'attention aussi du ministre-mais il le sait, je lui apprends rien. C'est que en cascade de tout ça. Il va y avoir un coût très important. Pour l'État. Parce qu'on est quand même dans une république. Il y a un pays qu'on aime et qu'il a quand même des spécificités et des garde-fous assez exceptionnelle par rapport à beaucoup d'autres pays. Même si il y a beaucoup à dire, mais quand même on reste quand même dans un certain niveau de protection donc au final. On va augmenter nos dépenses. C'est-à-dire qu'on va avoir c'est c'est ce ce paradoxe c'est qu'on va avoir de plus en plus d'hommes, de femmes voir d'enfants qui vont être privés de droits. Et on va augmenter la dépense publique. Pas augmentons peut-être la dépense publique mais au moins qu'elle soit source de droits nouveaux.

Merci. Il y a pas d'explication de vote que mais donc on voit cet amendement 29 avec 2 avis défavorable qui est pour. Qui est contre.

Merci monsieur le président. Hein conditionnant l'octroi des délais de paiement à la reprise des paiements de loyers et des charges avant la date de l'audience l'article quatre porte atteinte au dispositif de présomption des expulsions locatives. supprimant la suspension d'office par le juge de la Cour de résolutoire vous allez précipiter des des dizaines de milliers de personnes vers la solution. Cette mesure accroît inutilement la pression sur les familles en difficulté de paiement, dans un contexte économique et social particulièrement mal choisi pour fragiliser encore davantage les personnes les plus vulnérables. Couplé à l'accélération de la procédure d'expulsion prévue à l'article 5 elle empêchera les services sociaux. Les acteurs de solidarité de réaliser correctement leur diagnostic social et financier de mobiliser des aides pour trouver des solutions amiables et organiser la reprise des PMA. Notre groupe demande tout simplement la suppression de cet article. Nous pensons-nous cet article 18 que le la la demande en fait. De reprise du paiement de loyer. Avant l'audience a est excessive et elle est pas loyal en fait à l'égard des personnes en difficulté. Victime pour la quasi-totalité d'un accident de la vie, une perte d'emploi, une maladie et etc. Si un diagnostic social et financier doit être réalisé, nous constatons qu'une grande part des ménages arrive à l'audience. Sans avoir été convoqué par un travailleur social ou en n'ayant pas pu le rencontrer ou lit rencontré tardivement et brièvement. Ne sont donc pas informés, ni accompagnée assez tôt dans la mise en oeuvre d'aide ou de démarche. France aussi. Elle surendettement et cetera. C'est dû à la saturation des services sociaux qui n'est plus à démontrer. Avec le nombre de postes vacants et non remplacés. CAPEX les commissions de coordination des actions de prévention des expulsions. La Cour des comptes elles-mêmes constate qu'elles ne peuvent étudier qu'un nombre marginal de dossiers dont elle s'en saisisse. Même pas un petit c'est un ordre marginal et locataires ne sont donc pas informés, ni soutenu dans la reprise du paiement du loyer. Ce n'est d'ailleurs pas le réflexe 1er car le bailleur sollicitent avant tout le remboursement de la dette et a pu d'ailleurs parfois les paiements ultérieurs sur cette dette et non pas sur le loyer courant. Pour les bénéficiaires de. De l'allocation logement. Il est important d'avoir à l'esprit que c'est la décision de justice accorde un échéancier qui décidera la CAF à rétablir l'ordre, l'aide et donc aux ménages, leur permettra de reprendre le règlement intégral de leur loyer. Cet amendement a été rédigé en grande partie, je dois le signaler grâce aux travaux de la Fondation Abbé Pierre. Oui, merci Monsieur. Le président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, enfin sur les horaires, on se rappelle hein c'était une niche encadré par un temps. Et et le gouvernement a décidé que évidemment on y consacre tout le temps nécessaire pour que cette loi soit assurément voter. Voilà donc on est collectivement tous dans cette situation je en remercie de prendre acte de ça. Sur l'alinéa 4 de l'article 4. Alors là il y a une curieuse anticipation du jugement de rétablissement du bail du locataire alors il devra avoir remboursé l'intégralité de sa dette pour espérer avoir droit retrouver un logement de droit commun et bénéficier d'un bail en bonne et due forme. Bon on va continuer Ou lorsqu'ils sont en capacité de débloquer une aide comme le Fonds de solidarité logement par exemple. Donc ces jugements servent également de déclic à des personnes qui ont pu ne pas manifester de signaux positifs concernant le paiement du loyer, parfois pendant plusieurs mois ou plusieurs années et qui vont suite au jugement retrouver de l'espoir en bénéficiant d'un sursis dans leur processus d'expulsion ou d'un soutien pour retrouver un droit à l'APL. C'est notamment le cas lorsqu'un plan d'apurement et et mis en oeuvre avec l'appui d'un travailleur social, ce qui permet d'ailleurs beaucoup plus facilement d'obtenir un remboursement que lorsque vous enfoncer le clou avec une expulsion systématique sans solution de relogement derrière aggravant donc les possibilités d'insertion et de perception d'un salaire pour locataires en impayés en gros on va obliger à la fois les locataires à reprendre le paiement du loyer en amont et avoir remboursé la dette locative. je pense que ce mécanisme va dégrader la situation d'énormément de gens, voilà, c'est le sens de cet amendement. Très bien. Ensuite, nous avons encore 2 amendements identiques dans cette série. Celui de monsieur Ben Roche le 19 et celui de 31 ans suivent de monsieur Savoldelli. Dans le même article entre alinéa qui va dégrader la situation c'est l'alinéa 5. Supprimer la suspension de la clause résolutoire d'office par le juge en fait. Va précipiter des dizaines de milliers de personnes vers l'expulsion. Nombre de personnes que ni les services de prévention des expulsions locatives ni l'offre de logement social, ni les capacités d'hébergement complètement saturé ne pourra en aucun cas être en capacité d'absorber en peine déjà je vous le rappelle. À reloger les ménages Dalo. Le locataire doit scrupuleusement respecter l'échéancier qui lui est fixé, en plus de payer mensuellement sur loyer sur quoi le bail résilié. Donc le bailleur n'est aucunement lésés. La décision de justice est respecté. Il est payé et sur locataire reste elle ne l'est pas et la discussion a lieu. Il faut prendre en compte que cette disposition de suppression de la suspension de clauses réseau du soir s'ajoute aux autres mesures de la loi, déjà très sévère et préjudiciable pour les ménages en a payé. La réduction des délais en amant la réduction des délais pour quitter les lieux. Une lourde amende s'reste dans le logement après décision de justice prononçant leur expulsion. La grande majorité des à payer de loyer intervient, je l'ai dit tout à l'heure, suite à des accidents de la vie qu'on permette au moins aux locataires qui en a la capacité de rester dans leur logement. Merci, cher collègue, Monsieur Savoldelli défend ou Madame. Lienemann des. C'est exactement le même. Amendement avec la même explication. On rit insiste lourdement les propriétaires ne sont pas lésés. Puisque le le locataire est obligé de payer son loyer. Selon l'échéancier qui a été défini. S'il le fait il peut rester dans les lieux. S'il ne le fait pas. L'expulsion a lieu donc franchement je ne vois pas la nécessité de de mettre encore la tête sous l'eau supplémentaire à des gens qui ne sont pas tous des mauvais. Payeurs des gens irresponsables complètement mais parfois des gens dans une détresse sociale ponctuel et au contraire, tout doit être fait dans la société pour leur permettent de rebondir et de retrouver un chemin normal. Merci monsieur le président. C'est un peu un amendement de repli. Qui consiste à donner une garantie d'accès supplémentaire à un droit qu'une partie des justiciables peut ignorer. Étant donné que le bailleur et le locataire peuvent déjà. Saisir le juge a fait de suspendre les effets de la clause de résiliation de plein droit, comme le précise l'article 4 de cette proposition de loi. Nous demandons à ajouter la possibilité d'auto-saisine pour le juge. Pourquoi. Parce que cette demande que nous faisons, découlent de la méconnaissance. De certains justiciables de leurs droits, puisque les locataires dans la précarité manquent souvent d'information sur leurs droits et sur les modalités pour les actionnaires peut me dire qu'on va faire en sorte d'améliorer et cetera. La formation voilà bon mais en attendant d'améliorer la formation. Et étant donné que la connaissance des droits est essentielle, puisqu'elle permet à l'individu, de savoir ce qui lui est dû. Ou ce à quoi il peut aspirer et étant donné que le droit peut s'avérer difficilement compréhensible. Tout le monde le sait, y compris ici voire inaccessible pour les justiciables. Qui ne connaît pas forcément les procédures. Je ne vois pas en quoi le fait que le juge puisse s'autosaisir. Serait préjudiciable à quiconque. On peut en lui permettant de se se saisir lorsqu'ils le pensent nécessaire en fait c'est la seule garantie d'accès au droit de suspension avec l'égalité et l'équité de chacun devant la loi soit effective depuis. Nous estimons que le juge ait un arbitre. Et sa qualité de professionnel garanti une impartialité une compétence pour juger correctement de la nécessité de s'saisir. Dans la mesure où le droit et notamment la législation au droit immobilier est particulièrement complexe, nombreux sont ceux qui ne savent pas qu'ils peuvent sanctionner a-t-elle levier alors tout à l'heure, on n'a pas fait confiance à l'État ne fait pas confiance aux préfets. En fait pas confiance au juge. La confiance à quoi en fait uniquement au droit de propriété. Voilà les 6 amendements était présenté monsieur le rapporteur. Vous avez à donner l'avis de la commission sur les six. Ce président, Monsieur le Ministre, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, comme je l'ai exprimé tout à l'heure en discussion générale. C'est cet article IV qui a constitué le principal point de désaccord entre l'Assemblée nationale et le Sénat. L'Assemblée nationale. Ne souhaitait rappelez-vous initialement supprimer intégralement les pouvoirs d'office du juge en matière d'octroi de délais de paiement de vérification des éléments constitutifs de la dette locative du contrôle de la décence du logement et même de la suspension des effets de la clause résolutoire c'est-à-dire le maintien dans le logement. Cette suppression, rappelez-vous des pouvoirs d'office du juge nous est apparu ici au Sénat. Aussi bien pour des raisons évidentes pour le locataire. Et pour le bailleur. En effet le maintien dans le logement doit être privilégié pour inciter le locataire en difficulté à régler sa dette locative selon un échéancier d'apurement de la dette établie selon nous par le juge. lors de la première lecture nous avons rétabli les pouvoirs d'office du juge sur tous ces points en conditionnant cependant à la reprise du versement du loyer courant par le locataire. Ce qui nous semble une condition minimale afin de satisfaire le bailleur et de responsabiliser le locataire qui se doit d'honorer ses engagements contractuels. Nous avons en parallèle et on l'a dit déjà ici. Ajouter des dispositions permettant de rendre plus précoce. L'élaboration du diagnostic social et financier et d'accroître les pouvoirs des fameuses CAPEX hein. Commission de coordination des actions de prévention d'expulsion dans l'optique de mieux accompagner les locataires les plus en difficulté sans que cela soit à la charge des bailleurs. que mes chers collègues. Ces points ont nécessité d'âpres négociations avec le rapporteur de l'Assemblée nationale, qui est également l'auteur de cette proposition de loi et nous sommes parvenus à une rédaction de compromis qui tient compte des lignes rouges du Sénat les pouvoirs d'office du juge ont été en grande partie rétabli. Grande partie rétabli. Nous pouvons donc nous satisfaire de cette. Rédaction j'aurais aimé qu'il soit totalement établi. Nous pouvons donc nous satisfaire de cette rédaction que je vous invite à à voter conforme.

je veux redire et pour terminer ce ce travail. Que. L'expulsion locative est un échec pour un locataire de bonne foi en difficulté c'est pour ça que le travail que vous avez menée qui renforce la CAPEX et qui aux fruits des échanges comme la rapporte dit monsieur le rapporteur. Sur cet article 4 donne un, un résultat équilibré qui continue évidemment à préserver le pouvoir du juge d'abord le pouvoir du juge d'apprécier la reprise des paiements. Avant. L'arrivée en justice et puis en présence. Du locataire en en difficulté ou son représentant en en séance pourra accorder accorder des délais donc les pouvoirs du juge sont maintenues. La position d'équilibre entre l'Assemblée. Et le Sénat a été trouvé et donc je souhaite le maintien du texte en l'état et donc défavorable à cet amendement. Merci. Monsieur Bénard Roche souhaite expliquer son vote. Oui, monsieur le Président, puisqu'on a un peu d'avance. le rapport quand vous avez très bien défendu. En fait ce que vous auriez pu. Valider c'est-à-dire l'amendement qui vous a été présenté, alors. Faire et défaire c'est toujours travailler. Le Sénat assez et en l'occurrence il avait bien c'est L'Assemblée nationale a défait. Ce que 12 mandat au Sénat, c'est de refaire et d'heure faire bien. Voilà donc c'est pour ça que j'attendais un avis favorable. Y a-t-il d'autres explications de vote sur ces six amendements. Si ce n'est pas le cas. Il nous reste un petit crédit pour respecter le souhait de monsieur Roche. Mais il y a les explications de vote sur le texte donc je mets aux voix l'amendement fait de monsieur Bois-d'avec 2 avis défavorable qui est pour. pour. Abstention je l'vois pas il n'est pas adopté le 18 et le 30. Est-ce que c'est le même vote. Le 19 et le 31, je suppose qu'il en va de même et enfin le 14. Même Gaudi. Aucun d'eux n'est adoptée. J'en viens donc à l'article quatre que je mets aux voix qui est pour l'article 4. Qui est contre. y a-t-il des abstentions il était adopté. Les autres dispositions de la proposition de loi ne sont pas en 2ème lecture mais donc mettre aux voix l'ensemble de la proposition de loi qui souhaite expliquer son vote. Une fois, deux fois Madame Estrosi Sassone. Merci, monsieur le Président, je voudrais dire combien notre groupe se réjouit de l'adoption définitive cette proposition de loi qui a conservé. Donc la plupart des apports qui ont été ceux du Sénat en première lecture et qui sont restés à l'issue à l'issue de l'examen en seconde lecture à à l'Assemblée nationale. Je pense que on l'a dit à plusieurs reprises mais on a véritablement trouvé à travers ce texte de loi, un point d'équilibre entre plus de fermeté contre les squatters et contre les locataires de mauvaise foi mais aussi en prévoyant une meilleure prévention des expulsions et donc un meilleur accompagnement des locataires dont on se garde bien de faire un quelconque amalgame. Avec des squatters ou avec des locataires de mauvaise foi, s'agissant de locataires de bonne foi qui peuvent rencontrer un certain nombre de difficultés mais je crois que ce soir et c'est très important. Nous envoyons aussi un signal très fort à l'endroit des propriétaires. Monsieur. Ah il souhaite expliquer son vote. Merci, monsieur le Président, je tenais simplement déjà à remercier toutes les personnes qui se sont. Investis dans cette proposition de loi qui vise à protéger les logements contre l'occupation illicite. Ah 1er lieu évidemment notre rapporteur mais également l'ensemble de la commission des lois. Monsieur le président. Un buffet, merci. Pour cet investissement. Vous savez comme moi que ce texte non seulement vise à clarifier le régime judiciaire du squat d'une part, mais il permet également d'accélérer le contentieux locatifs. D'autre part, le gouvernement n'a eu de cesse tout au long du processus législatif de je reprends vos propos, Monsieur le Ministre de d'équilibrer cette proposition de loi. Notamment lorsque vous avez dit que on ne devait pas réagir de la même manière contre les squats en particulier sont entretenus par des marchands de sommeil que devant les impayés des locataires au regard de ces différents arguments notre notre groupe votera pour cette proposition de loi. Nous allons pouvoir passer au vote sur l'ensemble du texte et j'ai été saisi sur ce scrutin d'une demande de scrutin public par le groupe RDPI. Je rappelle que. Nous sommes donc dans le vote final il va être procédé au scrutin public dans les conditions de l'article 56 du règlement. Le scrutin est ouvert.

personne ne demande à voter Le scrutin est donc clos. Voici le résultat du scrutin. Nous étions 343 votants. 339 exprimé pour la proposition de loi 248 contre 91. Elle est donc adopté. Monsieur le Ministre vous pouvez dire un mot. adoptée est équilibrée grâce au travail de l'ensemble des parlementaires et et vraiment. En mon nom je tiens et du gouvernement. Je tiens à vous remercier, remercier l'ensemble des séances que la qualité des échanges. Ce soir et et lors des 2 Lecteurs, Turow au Sénat ont montré l'importance que revêtait pour nous la question du, du logement et en particulier cet équilibre entre propriétaires et locataires et la manière dont on était attentif aux plus fragiles, mais aussi aux propriétaires et et je crois une forme d'unanimité sur. Le sujet des squats qui est effectivement un insupportable et et sur lequel nous devons lutter en particulier lorsqu'il s'agit de de marchands de sommeil et et j'en profite pour saluer. Guillaume Kasbarian qui a dû suivre nos échanges. Sur, sur Internet et et encore une fois, un grand merci et comme je suis pas tout à fait Cendrillon et qu'il est presque minuit. Très vite merci. Voilà, mes chers collègues, je vais lever la séance prochaine séance demain jeudi à 10h 30 pour les gamins de l'octroi des pouvoirs de commission d'enquête à de commissions. Puis pour l'examen de la PPL visant à assurer la pérennité des établissements de spectacle cinématographique et l'accès au cinéma dans les outre-mer la séance est levée.